Madame la Ministre, mes chers collègues, la séance est ouverte. Le compte rendu analytique de précédentes séances. C'est distribué pas d'observation, le procès verbal est adopté sous les airs d'usage. L'ordre du jour appelle l'examen de 2 projets de loi tendant à autoriser la ratification l'approbation de conventions internationales pour ces 2 projets de loi, la conférence des présidents retenu la procédure d'examen simplifiée. Je vais donc les maîtres successivement, au revoir. Je mais on voit le texte adopté par la commission sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après l'engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et la Cour pénale internationale sur l'exécution des peines prononcées par la cour, la commission des Affaires étrangères est favorable à l'adoption de ce texte qui est pour. Vous n'êtes pas nombreux mais si vous pouviez lever le doigt. Voilà qui est pour. Qui est contre. Très bien. Le projet de loi est adopté définitivement, je mais on voit le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement, la principauté d'Andorre relatif à l'exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatiques consulaires techniques et administratifs des missions officielles. La commission des Affaires étrangères favorable à tour de ce. C'est ce qui est pour. Voilà qui est contre. Voilà le projet de loi est adopté, si tout pouvait être aussi rapide. Allez hein. L'ordre du jour appelle la discussion en 2ème. Lecture de la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale, créant une aide universelle d'urgence pour les victimes des violences conjugales dans la discussion générale. La parole est à madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de la diversité et de l'égalité des chances. Vous avez la parole madame la Ministre. Monsieur le président. Madame la présidente de la commission des affaires sociales. Madame la rapporteure mesdames les sénatrices et les sénateurs. Nous tenons entre nos mains un objet précieux. L'un de ces objets législatif particulier qui, dès la seconde même où ces dispositions seront appliquées changera immédiatement des vies. Parce qu'en cas de violences conjugales. Il est toujours difficile de tourner définitivement le dos à son bourreau. Nous devons faire en sorte que lorsqu'une femme décide de recouvrer une liberté qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Rien ne puisse freiner son courage. Le drame de celles qui subissent au quotidien la violence de leur conjoint connaîtra grâce à cette proposition de loi, un facteur contraignant en moins. Bien sûr si je le pouvais si nous le pouvions nous de Riom chaque victime de violences physiques ou psychologiques. Nous ferions disparaître cette emprise mortifère par lequel les hommes violents détruisent à petit feu leur compagne si je le pouvais. Si nous le pouvions nous est de Riom chacune. De ses victimes à boucler sa valise. Ce que nous pouvons faire en revanche. C'est agir en acteur responsable des politiques publiques. C'est ce que fait le gouvernement via le Pack nouveau départ annoncé par la Première ministre dès septembre 2022. la sénatrice Valérie Létard. Merci madame la sénatrice, en déposant cette proposition de loi et c'est ce qu'on fait. L'Assemblée nationale et le Sénat en adoptant à l'unanimité ce texte en première lecture. Je suis convaincu que ce texte que vous examinez aujourd'hui en seconde lecture fera à nouveau l'objet d'un vote favorable et transpartisan. Je m'en réjouis de tout coeur. Face à ce fléau. Seule l'union fait la force. C'est pour que ce dispositif convienne à toutes et s'adapte à chacune. Quel que soit son parcours, son âge, son orientation sexuelle, son lieu d'habitation. Son statut social ou sa profession que le gouvernement a souhaité modifier l'article 1er de ce texte. Les principes énoncés dans cette proposition de loi sont ceux qui sont portées au dans notre République. Ce dont vous représentant du pouvoir législatif, être les gardiens. Ainsi, nous l'avons élaboré de manière à ce que, à ce qu'elles ne contiennent rien d'autre que des solutions pratiques qui permettent aux femmes une aide concrète au départ. Tout au long de ma carrière de magistrate, j'ai croisé des femmes. Qui n'était plus que l'ombre d'elle-même. J'ai écouté leurs souffrances des heures durant. J'ai dû juger arbitré. Apporter une réponse pénale à leur calvaire. Je me souviens. De Gisèle séquestré, violé pendant des mois chez elle par son conjoint. Qui, un jour, avec la complicité d'une amie par 20 à prendre la fuite de Solange qui par 20 à partir à à 75 ans. Après des années. D'humiliation et de violence. J'aurais voulu leur offrir bien plus mais ce n'était pas mon rôle. Alors. J'ai gardé leurs mots en mémoire. Et je n'oublierai jamais non plus les visages de celles que je n'ai vu que sur photo. Parce que c'était trop tard. Comme il a. Massacré toute la nuit par son conjoint, devant ses trois enfants. J'aurais voulu aider Leila à partir. Ces femmes. M'accompagne chaque jour. Particulièrement aujourd'hui. Cette proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui permettra à d'autres Gisèle Solange Leila de relever la tête de recouvrer la dignité dans leur bourreaux les à spolier. Chaque cas est unique, il nous faut apporter une solution même aux cas les plus complexes. Lorsqu'elle sera votée, cette proposition de loi viendra donc compléter et renforcer nombre de mesures que nous avons mis en place comme par exemple le Pack nouveau départ que j'ai proposé à la Première ministre, qui a été annoncé par elle-début septembre et qui vise à proposer aux victimes à parcours un parcours coordonné afin d'assurer le déblocage rapide de toutes les aides auxquelles elles peuvent prétendre et dont le président de la République a réaffirmé le caractère prioritaire le 25 novembre dernier. Je pense également au Grenelle. Auxquels j'ai activement participé lorsque j'étais au ministère de la justice et dont la quasi-totalité des mesures ont été mises en oeuvre grâce à vous, nous irons encore plus loin. Selon sa situation une femme victime de violences peut faire face à une multitude d'obstacles qui constituent autant de freins à son départ. Lorsque ces Opta peuvent être levées par des politiques publiques. Il est essentiel que nous soyons au rendez-vous. Car c'est aussi dans ce moment charnière que les victimes sont les plus faibles dans cette zone grise qu'elles ne connaissent que trop où tout peut encore basculer ou l'emprise trouve toute la place de s'exercer. Nous pouvons alors en faisant cesser cette situation de dépendance matérielle, économique, mettre fin à l'emprise et rompre le cycle de la violence. Car tout non départ tout retour en arrière peut être fatal. C'est pour cette raison que j'ai voulu que le prêt initialement prévue puissent aussi prendre la forme d'un don. Tout simplement parce qu'il est impensable que la victime se retrouve en position de débiteurs face à qui que ce soit du fait des actions qu'elle engage pour se protéger. Parce que le déséquilibre généré par un départ peut faire vaciller une décision déjà difficile à prendre et donc fragile et nous voulons à tout prix éviter un faux départ. Ce que nous proposons c'est de poser le principe d'une aide financière d'urgence aux victimes de violences conjugales. Cette aide sera financée par l'État et prendra la forme d'un don ou d'un prêt qui le cas échéant devra être remboursé par l'auteur condamné. Ce dispositif émancipateur lorsqu'il est attribuée sous forme de prêt aura le mérite de mettre l'auteur face à sa responsabilité financière. Il pourra dans le cas de la procédure pénale se voit réclamer le recouvrement de l'aide accordée à la victime. Nous faisons reposer notre proposition sur le triptyque de souplesse rapidité universalité souplesse parce qu'il nous faut. Répondre aux besoins de chaque victime rapidité parce que notre réponse doit prendre en compte chaque seconde passée en compagnie de son bourreau. Et que chaque set chaque seconde patients cette compagnie est une seconde de trop et universalité par ce que nous voulons que nos dispositifs soient accessibles sans conditions de ressources aux victimes qui en ont besoin. Vous l'aurez compris ce que j'appelle de mes voeux devant vous aujourd'hui, c'est que nous admettions ensemble que protéger nos concitoyennes du danger qui les guette dépasse les clivages partisans. En votant ce texte de loi vous permettez son application rapide en votant ce texte de loi vous soulager les souffrances de celle qui veut s'extraire des griffes de leurs bourreaux. Vous leur donnez le souffle pour partir vous sauver leur peau. Quel que soit notre appartenance politique nous devons vaille que vaille protéger ces femmes. À l'issue de cette séance, nous avons la possibilité de sauver des vies. Nous avons l'occasion de faire un pas de plus en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Saisissons-là. Merci, madame la Ministre, la parole est maintenant Madame Jocelyne Guidez, rapporteur de la commission des affaires sociales pour 10 minutes maximum. Monsieur le Président Madame la Ministre. Mes chers collègues. Le 20 octobre dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi créant une aide d'urgence en faveur des victimes de violences conjugales déposée par notre collègue Valérie Létard. Moins de 4 mois plus tard, le texte nous revient après avoir recueilli le vote là aussi unanime de l'Assemblée nationale il y a toutefois, qui a toutefois apporté des modifications substantielles. La proposition de loi adoptée par le Sénat prévoyait un dispositif d'avances d'urgence octroyées par les caisses d'allocations familiales sous la forme d'un prêt à taux zéro, l'objectif poursuivi par cette avance et d'aider les victimes à quitter le domicile conjugal alors que 19% des femmes victimes d'éclats subir des violences économiques lors de leur appel aux 39 19 Le 1er des 3 versements mensuels constituant c'était devait intervenir dans les trois jours ouvrés suivant la la demande. Le dispositif et ses paramètres étaient issus des retours d'expérience d'une expérimentation menée dans le nord par le conseil départemental et la Caisse d'allocations familiales. En outre, le texte que nous avions adopté assortissait c'est le service de l'aide d'un mécanisme de remboursement par l'auteur des violences conjugales. La CAF avait la possibilité de se constituer partie civile pour le compte de la victime si ça-ci a renoncé à exercer ses droits afin de récupérer les sommes sur les dommages et intérêts, prononcés lors d'un procès pénal. Nos collègues députés ont apporté au texte du Sénat des modifications qui ne sont pas négligeables. Certaines ont été portées par le gouvernement qui à cette occasion est sorti de la réserve dont il avait fait preuve devant nous. Toutefois, la proposition de loi à garder intact l'ambition de donner aux victimes de violences conjugales dans un délai très court, les moyens financiers pour se séparer du conjoint violent. C'est pourquoi la commission adopté cette profession de loi sans modification pour permettre son application rapide. L'article 1er du texte qui porte le dispositif de l'aide d'urgence a fait l'objet d'un amendement de rédaction globale du Gouvernement sous- amendé à de nombreuses reprises. Il faut souligner d'emblée les motifs de satisfaction du texte qui nous a été transmis. Le financement de l'aide d'urgence a été transféré de la Caisse nationale des allocations familiales à l'État qui assumera la une mission qui lui incombe naturellement l'Assemblée nationale a également affirmé le droit de toute victime conjugal à bénéficier d'un accompagnement global. Enfin, le gouvernement a pu proposer des modifications que nous appelions de nos voeux mais que les règles de recevabilité financière nous nous permettait pas de réaliser. Je ne par exemple, les caisses de la Mutualité sociale agricole se trouve désormais intégré au service de cette nouvelle aide, ce qui est nécessaire afin d'atteindre leur allocataires. Ce sont des caractéristiques de l'aide sa nature a tout d'abord été dédoublé avec la possibilité d'octroyer à la victime soit un prêt soit une aide non remboursable selon sa situation financière et sociale qui était très important. La détermination du montant de l'aide a également été revue le montant pourra être modulé, dans le respect de plafond limitatif selon l'évaluation des besoins de la personne notamment sa situation financière et sociale. De même le montant devra tenir compte de la présence d'enfants à la charge de la victime. Ce que nous avions souhaité au Sénat cette modulation semblait impérative, alors que dans la plupart des cas des victimes ne quitte pas le domicile sans leurs enfants. L'Assemblée nationale a également assoupli les délais de 1er versement de l'aide. Le délai pourra par dérogation est portée de 3 à 5 jours ouvrés. Dans le cas où la victime n'ait pas déjà enregistrées comme locataire de l'organisme payeur cet allongement n'est pas souhaitable en soi mais demeure plus conforme aux inquiétudes avancées par la CNAF et au délai qui pourront réellement être respecté par les caisses sur le terrain. Enfin, toujours à l'article 1er, le mécanisme de récupération de l'aide a été amendé en conservant le principe de demander le paiement à l'auteur des violences lorsque l'aide est versée sous la forme d'un prêt le remboursement fait partie des peines que les juridictions pénales peuvent prononcer contre l'auteur reconnu coupable ainsi que les dispositifs à la main des parquets. Dans le cas d'un classement sous condition de la procédure ou de mesures de composition pénale. La navette a donc enrichi l'article 1er de nouvelles dispositions. Toutefois, comme vous pouvez le constater, elle demeure fidèle à l'objectif du texte adopté par le Sénat. Nos collègues députés ont d'ailleurs maintenu inchangés les conditions d'octroi de l'aide d'urgence ainsi que le bénéfice au droit et à d'accessoires au RSA qui accompagne le versement de l'aide pécuniaire à l'article de. Les députés ont maintenu l'obligation faite aux gendarmes et policiers d'informer la victime déposant plainte de la possibilité de demander de l'aide d'urgence. En revanche, si l'enregistrement à la demande dans le commissariat ou la gendarmerie demeure une faculté, elle n'est plus systématique. Sans doute. Les députés ont-ils estimé que de telles dispositions ne serait pas appliquée par la norme contraignante mais par les engagements volontaires des acteurs du terrain. D'autres dispositions de la proposition de loi concerne son appui qu'habilités aux outre-mer comme vous le savez, mes chers collègues, en profession les victimes de violences conjugales sont encore plus nombreux en outre-mer que dans l'Hexagone. L'article 1er bis habilite ainsi le gouvernement à légiférer par ordonnances pour adapter la loi à Mayotte. Enfin, l'Assemblée nationale a inséré quelques nouveaux articles pour avoir examiné ces dispositions commissions la sincérité m'oblige à dire que leur pertinence est toute relative, mais ces dispositions sont annexe au dispositif de l'aide d'urgence et ne gênent pas son application. L'article 1er terre propose ainsi que nos lois de programmation pluriannuelle détermine la trajectoire des finances publiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes pour symbolique et médiatique que soit cette disposition, elle est dépourvu de portée normative. Le gouvernement ne pouvant constitutionnellement, être tenus de déposer un tel projet de loi. Enfin, les articles de terre et de quater sont des demandes de rapports sur lesquels une fois n'est pas coutume, la commission a été indulgent. En 2ème lecture. La commission a donc adopté sans modification le texte transmis en raison du maintien de l'essentiel de la proposition de loi adoptée adoptée par le Sénat et des améliorations introduites par la navette parlementaire. Nous nous réjouissons, notamment de la suppression de l'article 3, par un amendement du gouvernement permettant ainsi de lever le gage financier une n'adoption conforme du texte aujourd'hui signifierait une belle avancée d'initiative sénatoriale dans la lutte contre les violences conjugales issu de l'expérience de nos territoires. Cette proposition de loi qui entrera en vigueur au plus tard 9 mois après sa promulgation, viendra utilement compléter les dispositifs existants. C'est pourquoi la commission vous invite à adopter la proposition de loi dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est maintenant à madame la présidente Laurence Rossignol. Pour le groupe socialiste pour six minutes.

Monsieur le président, madame la ministre madame la rapporteure monsieur le vice-président de la commission. Je suis d'abord. Je voudrais renouveler à notre collègue Valérie Létard nos remerciements. pour sa rédaction pour le dépôt de cette proposition de loi pour son obstination et l'énergie qu'elle a mise à la faire adopter la vigilance qu'elle a exercée sur le parcours du texte et me réjouir aujourd'hui que cette proposition de loi soit adoptée, il est temps que la navette parlementaire s'arrête que le texte soit adopté promulguée et mise en oeuvre. Les femmes l'attendent et nous avons là un bon texte, je crois que nous allons déboucher aujourd'hui l'un des premiers écueils à la dénonciation des violences subies. Et la crainte de devoir quitter le domicile et de se retrouver sans ressources dans une précarité matérielle et qui pose une question de survie quotidienne. Et cette crainte est d'autant plus grande, et a cru que la femme a des enfants à charge. Et cette crainte peut être suffisamment forte peut si forte que les femmes ne vont pas demander d'aide, elles ne vont pas dénoncer leur calvaire. Elles ne vont, à rester au domicile conjugal domicile conjugal qui est désormais pour elle une prison où les enferme l'auteur de ces violences. C'est notamment pour cette raison que la défense de l'indépendance économique des femmes, plus globalement. Est crucial. C'est une étape indispensable dans l'émancipation que les femmes soient ou non victimes de violences. Nous avons progressé à grands pas sur le sujet. Grâce aux mobilisations féministes accès au compte bancaire doit travailler sans le consentement du mari, suppression des interdictions professionnelles faites aux femmes et caetera et caetera. La liste est longue et réjouissante. Nous poursuivons cette mobilisation à travers différentes initiatives pour avancer sur le chemin de l'égalité professionnelle, faire tomber les stéréotypes qui entravent l'orientation des filles et en cette journée consacrée au numérique. Je souhaite attirer l'attention du Sénat sur la faible part de femmes dans le numérique dans ces métiers de demain qui nous prive d'un nombre d'ingénieurs important si les femmes si à s'engager dans ces métiers qui prive ce secteur. De ressources humaines et qui prive les femmes d'accès à des métiers qui seront demain des métiers importants. Dans ces mesures que nous devons encore prendre pour éliminer les inégalités salariales accompagner les mères monoparentales défendent l'augmentation des bas salaires. Nous avons déjà des outils et je c'est pour ça que je défends régulièrement quelques propositions comme la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial ou encore l'augmentation du SMIC, puisque je rappelle que 160% des salariés au SMIC sont des femmes. Augmenter le SMIC, c'est augmenter les salaires des femmes. Mes chers collègues, nous fêtons cette année les 5 ans du mouvement MeToo, grâce aux témoignages grâce au mouvement féministe grâce à la mobilisation d'associations et de l'ensemble de la société grâce à la mobilisation des pouvoirs publics et j'ajouterai maintenant grâce à la mobilisation des collectivités locales qui est un élément nouveau dans la lutte contre les violences. Intrafamiliales j'ai observé d'abord cette année au congrès des maires de France, un atelier était consacré. Nous y étions Madame la Ministre. À la manière dont les collectivités locales pouvait s'impliquer et je vois sur le terrain dans mon propre département que c'est un sujet en lien avec la gendarmerie, d'ailleurs le plus souvent des délégués Droits des femmes dont les collectivités locales les EPCI s'empare, qu'est-ce qu'on peut faire comme entrée comment apporter une réponse 3 types de violences conjugales concerne collectivités locales, celles dont sont victimes les habitantes de leur de celle dont sont victimes les salariés, les fonctionnaires territoriales dans leur commune ou leur collectivité locale et enfin celle subie par les conseillères municipales et les élus et sujet parfois plus difficile, celle effectuée par des collègues conseillers municipaux. Malheureusement, les statistiques globales ne sont pas différentes dans chaque catégorie, chaque échelon de la société nous retrouvons strictement les mêmes. Mais je trouve que cette mobilisation des collectivités locales est un élément fort important et tout à fait. Encourageants pour éradiquer les violences faites aux femmes. voudrais pas. Trop 10 graissé mais nous avons encore beaucoup de chantier la restriction des modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement. L'exclusion de la résidence principale de l'enfant chez l'auteur de violences, l'augmentation de la durée de la portée des conditions d'accès à l'ordonnance de protection. La dissimulation d'adresse de résidence et de l'école des enfants au à à l'ex-conjoint violent. Le signalement à la victime de la remise en liberté de son agresseur présumé, le renforcement de la lutte contre les violences et de peu séparation l'abrogation du délit de non-. Représentation d'enfant qui est une arme à fragmentation contre les femmes aujourd'hui contre les maires qui protègent leurs enfants et enfin le très beau chantier Madame la Ministre dont je connais. Votre engagement pour lequel je connais votre engagement votre volonté d'aboutir, de réussir et aux côtés, nous serons à vos côtés pour le faire, celui de la mise en place d'une justice d'une juridiction spécialisée en matière de violences intrafamiliales conjugal et sexuel qui rassemble justice civile et justice pénale la création d'une aide financière d'urgence hein sont des victimes et donc un moyen concret immédiat ça ne résout pas tout, mais c'est essentiel ce que vous avez proposé aujourd'hui madame chère collègue Valérie Létard. Je voudrais dire enfin tous les la violence les violences contre les femmes coûte 3,3 milliards d'euros par an à la société et que donc les sommes que nous allons engager par l'intermédiaire des caisses d'allocations familiales sont bien peu comparé au coût collectif que nous assumons, du fait de ces violences. Je vous remercie, cher collègue. Merci cher collègue là. La parole est maintenant à madame Laurence Cohen pour le groupe CRCE pour 4 minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre Madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales que nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture aura connu un parcours les plus tumultueux cette proposition de loi de notre collègue Valérie Létard reprenait une proposition de loi déposée par ma collègue Michel Legré, homme en février 2021. Je veux les en remercier, ainsi que notre rapporteur Jocelyne Guidez. Face aux nombreuses insuffisances de l'action publique en matière de lutte contre les violences conjugales. Le gouvernement a déposé et fait adopter un amendement visant à réécrire intégralement l'article 1er. Nous saluons le fait. Que Que plusieurs amendements GDR nos homologues à l'Assemblée nationale ait été adopté pour encore enrichir le texte et supprimer la condition que le gouvernement avait instauré sur la régularité au séjour et sur les difficultés financières immédiates une aide universelle se doit de l'être, même si elle est modulée en fonction des besoins. Le fait que la présence d'enfants à charge ait été pris en compte et que ce soit l'état et non plus la CNAF qui gère ses dépenses de l'aide sont également des mesures positives. L'introduction de l'article 1er terre qui prévoit une loi de programmation pluriannuelle de lutte contre les violences faites aux femmes, en ciblant l'accompagnement psychologique et social, l'hébergement, la formation est extrêmement importante. Madame la Ministre même son caractère normatif, pouvez-vous nous confirmer que cette loi verra le jour avec les moyens nécessaires, que cela soit pour le 39 19 comme cela d'ailleurs est prévu, comme pour l'ensemble des associations qui nous alertent les groupes LR et centristes à l'Assemblée nationale ont également enrichi cette PPL et si j'ajoute enfin que plusieurs amendements du groupe socialiste ont complété le texte, en précisant notamment que l'accord de la victime était nécessaire avant l'information du président du conseil départemental, vous aurez la un texte largement transpartisan cette construction partagée s'explique en grande partie par la progression des violences conjugales dans notre pays, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes 113.000 femmes ont été victimes de violences physiques et sexuelles commises par leur partenaire ou ex-partenaire en 2019. Le ministère de l'Intérieur par a fait paraître une alerte sur l'augmentation de 20% en 2021 par rapport à 2020 du nombre des féminicides 122 de nos soeurs, nos mères, nos cousines nos voisines, nos filles, nos amis sont décédées sous les coups d'un conjoint ou ex- conjoint, contre 102 en 2020. Par conséquent, il est indispensable d'accompagner les victimes de violences conjugales à sortir de l'emprise morale économiques exercées par le conjoint l'instauration d'une aide financière d'urgence aux victimes permettra donc d'encourager cette démarche de départ salvatrice. Nous ne pouvons que regretter Madame la Ministre permettez-moi de revenir là dessus que la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron ne bénéficient pas des 2 milliards d'euros qui sont demandées par les associations féministes afin d'engager une lutte véritablement efficace contre les violences en agissant sur l'éducation et la prévention plutôt que d'attendre l'apparition des comportements violents. je vais profiter de ce moment pour insister Madame la Ministre sur un fait important si nous voulons et je sais que c'est votre objectif, débarrasser notre société de ce fléau. Je vous appelle à soumettre au Parlement assez rapidement un projet de loi cadre sur les violences faites aux femmes, en vous appuyant sur le travail. Qui est fait par les associations féministes et notamment le collectif national des droits des femmes. C'est mon souhait, c'est notre souhait, je crois que nous ne partageons en attendant les sénatrices et sénateurs de mon groupe, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste votera favorablement ce texte en espérant une adoption conforme pour une entrée en vigueur le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci cher collègue là. La parole est maintenant à la présidente Valérie Létard pour le groupe Union centriste pour six minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre. Monsieur le Président commission madame la rapporteure, chers collègues. Nous voici arrivés à la fin du processus d'examen de la proposition de loi sur l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales que j'ai souhaité, avec l'aide de mon groupe porté au débat devant le Parlement et. Dans un délai record Laurence Rossignol la signalé en madame la rapporteure aussi en 4 mois à peine. C'est assez. Extraordinaire pour ce type d'exercice c'est forcément aussi avec un sentiment. Particulier une Particulier une émotion certaine sincère que je prends la parole pour exprimer. Un mélange de satisfaction de joie de fierté partagée. Qui m'ont par. À ce moment de nos débats. Qu'une initiative de terrain. Qui s'est construit grâce, un travail nourri par les professionnels de mon territoire à l'expertise de nos administrateurs qui ont su à travers d'échange d'expériences d'expertise traduire une volonté d'aboutir à un texte. Adapté à la réalité quotidienne que vivent les professionnels dans leur action auprès des victimes de violences. Et bien évidemment aussi trop souvent de leurs enfants. Un texte qui je l'espère, nous l'espérons tous contribuera à changer la vie et le destin de nombreuses, de trop nombreuses victimes sous emprise grâce à une aide financière qui devra être simple d'accès, et dont le montant et les modalités Madame la Ministre devront au travers au travers du décret que vous avez la la grande responsabilité de mettre en oeuvre. Être à la hauteur des besoins. Une aide universelle qui pourra prendre la forme d'une aide non remboursable ou d'un prêt partiellement ou totalement remboursable, vous en avez changé les mots. Madame la ministre, en remplaçant cette notion de prêts bénéficiant de remises totales ou de réduction en une, un, dont une aide non remboursable ou un prêt. Sans intérêt. Le but, vous en conviendrez, est le même, c'est un soutien financier ambitieux accessible rapide et lisible, facile d'utilisation par les professionnels permettant de libérer de l'emprise financière de leurs bourreaux. Celles et ceux qui en sont victimes. Bon dans cette période de répète pendant une période nécessaire pour rétablir les droits de ceux qui les ont perdu de cette absence de financement dans l'urgence, il n'y a pas de classe, pas de milieu, pas de génération. Pas de situation socio-professionnels, qu'ils soient épargnés par cette triste réalité des violences au sein du couple l'universalité était donc essentiel à mes yeux, à nos yeux. Peut-on exclure une femme salarié privé de ses propres ressources une jeune de moins de 25 ans qui a pas droit au RSA, une personne retraitée. Non. Et donc ce dispositif imaginé universel et rapide. Ah visant à n'exclure aucune victime. Quelle que soit sa réalité était indispensable. Merci madame la rapporteure. Merci aussi à Monsieur le Président vous ça durée aussi, madame la présidente pour l'écoute attentive qu'a eu la commission et bien évidemment si nos collègues pour entendre nourrir, enrichir des amendements divers de l'investissement de nos collègues sur ce texte. Votre écoute vous avancez n'ont fait que renforcer encore la portée de ce texte notre unanimité en première lecture a été inspirante et a permis, je pense au gouvernement Madame la Ministre hé bien de changer la position des partis était plutôt réservé et de vous donner la possibilité d'aller plus loin. L'Assemblée nationale et on peut remercier aussi la présidente de l'Assemblée qui a su créer les conditions d'un examen transpartisan. Et un vote unanime après des modifications apportées par les rapporteurs et je salue ma collègue, Béatrice Descamps, qui était rapporteur et qui est ma collègue du Nord. Les différents groupes aussi de l'Assemblée, vous l'avez dit, Madame Cohen ont apporté et nourrit ce texte et ils ont réintégré des dispositions qui n'étaient pas toutes dans la position et dans la l'amendement du gouvernement. Cela permet d'avoir rajouté l'accompagnement social et professionnel. Les droits sociaux liés qui sont indispensables, une transmission de la demande simplifié à la CAF et au département et aussi, madame la ministre vous remerciez évidemment d'avoir maintenu la possibilité de se retourner sur l'auteur des violences pour le remboursement ou encore d'avoir levé des gages pour la familialisation et et possibilité aussi donner à la MSA de gérer ses propres ressortissants. Unanimité au Sénat et à l'Assemblée, ceux-là montrent que même dans les périodes de tensions l'intérêt général et la portée des sujets tels que celui qui nous réunit transcende les courants et montre le sens des responsabilités de nos assemblées. C'est un bel exemple dans les moments que nous vivons. La loi doit protéger les plus fragiles d'entre nous ce principe essentiel m'a toujours guidé et si vous êtes là, à cet instant et si vous tenez ces propos c'est bien parce que vous le partagez et que vous le défendez tout autant que moi et je vous en remercie. Merci à vous tous et j'en arrêterait là de donner tout son sens à l'engagement politique et à l'action publique. Car ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une vraie avancée et c'est pour cela je pense que toutes et tous, hé bien toujours été mobilisés déterminés à faire avancer la cause des plus vulnérables avant tout le destin de notre pays, sans laisser personne au bord de la route nous pouvons. On être collectivement très fier. Merci à toutes et à tous. La parole est maintenant monsieur Éric Gold pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Excusez-moi je remets de l'ordre dans ma chemise. Merci monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente. De commission madame la rapporteure, chers collègues. 4 mois après l'adoption de cette proposition de loi à l'unanimité. Nous nous retrouvons donc pour examiner le texte en 2ème lecture après son adoption à l'Assemblée nationale, à l'unanimité également. Mais avec plusieurs modifications. Si ces modifications ont fait craindre un report dans l'application de la mesure. Elles ont néanmoins permis d'améliorer le texte, notamment grâce à l'engagement du gouvernement sorti de sa réserve initiale. Sur un sujet aussi majeur que les violences conjugales. Nous pouvons saluer le travail consensuel effectués au sein du Parlement et de l'exécutif. Quand il s'agit d'aider les victimes à s'extirper des nains de leur bureau de leur bourreau. Nous sommes heureusement capable de travailler en bonne Intelligence. Près de 300.000 personnes sont victimes chaque année de violences conjugales en France, 72% d'entre elles sont des femmes. Or il est avéré que la précarité financière retarde, voire empêche le départ du domicile conjugal et on ne sait que cette. Précarité touche davantage les femmes. En complément des aides déjà existantes. Je rappelle le téléphone grave danger le bracelet anti-rapprochement et toutes les mesures du Grenelle des violences conjugales. Cette proposition de loi s'attaque donc spécifiquement à la question de la dépendance financière qui demeure un frein majeur pour nombre de victimes. Conservant l'esprit initial du texte. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale se décline en un prêt à taux 0 et une aide non remboursable modulée en fonction des besoins de la victime et de sa situation économique et sociale. La présence d'enfants à charge pourra notamment permettent l'octroi d'un montant supplémentaire qui devrait aider à les sortir de ce climat de violence dont ils sont aussi les principales victimes. Dans le cas d'un prêt et sur décision de justice le remboursement pour être mis à la charge de l'auteur des violences, ce qui libérera de fait la victime de sa créance. Cette aide est toutefois conditionnée à un dépôt de plainte ou un signalement au procureur de la République. Les commissariats et unités de gendarmerie pour enregistrer et transmettre la demande d'aide, sans y être obligée, seule demeure l'obligation d'informer la victime de l'existence de cette aide, ce qui semble en effet plus conforme au rôle et missions des forces de l'ordre. Hormis les articles qui sollicitent les demandes de rapport auquel nous sommes au sénat et au groupe RDSE généralement très réticents. Nous regrettons l'inscription du demande de loi de programmation pluriannuelle sur la trajectoire des finances publiques en matière de lutte contre les votes. Violences faites aux femmes. Elle n'a qu'une portée symbolique puisque le gouvernement n'est pas tenu de déposer un tel projet de loi. Gardons-nous de créer de faux espoirs en la matière. Enfin si la rédaction issue de l'assemblée correspond à la volonté générale des auteurs de la PPL de créer une aide universelle, la suppression de la condition de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France me paraît en réalité peu opérationnel chaque victime doit bien sûr pouvoir être aidé mais je doute que les personnes en situation irrégulière se rendent au commissariat pour porter plainte et je crois que nous devrions nous concentrer sur des aides plus adaptés à leur réalité. Pour conclure cette proposition de loi offre une aide supplémentaire dans cette période de latence que constitue le départ parfois brutal du domicile et sur le de sujets très complexes de la dépendance financière qui rajoute à la vulnérabilité repousse indispensable mise à l'abri si ce nouveau droit peut convaincre, ne serait-ce qu'une seule victime de partir alors. Nous aurons peut-être sauver une vie. De plus, le groupe RDSE votera donc comme en première lecture cette PPL d'une seule voix. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est maintenant à Madame Valérie Boyer pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.

Elles avaient 19 30 51 ou 90 ans la plupart était mère de famille, leurs enfants parfois été témoin de cette barbarie ou même été tués à leur tour. Certaines étaient enceintes. Parfois, elles ont été brûlés vifs poignardée étranglée ou abattu d'un coup de fusil ces meurtres perpétrés sur tout le territoire français sans. Seulement par des hommes qui étaient déjà parfois connu des services de police et même souvent et de la justice. Six pour des faits de violences conjugales en 2022, 147 d'entre elles ont été tuées par leur conjoint et ex-conjoint et je voudrais souligner que 18 hommes aussi ont été tuées par leur conjoint ou leur conjointe. Un enfant est tué par l'un de ses parents, tous les 5 jours en moyenne, d'après l'UNICEF. Près de 400.000 enfants en France vivent dans un foyer où les violences intrafamiliales sévissent derrière chiffre il y a une réalité, celle de la souffrance insupportable et inacceptable. Plus jamais, plus que jamais par dont nous avons besoin de la. Application de tous. C'est pourquoi le 20 octobre dernier, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi créant une aide d'urgence en faveur des victimes de violences conjugales déposée par notre collègue Valérie Létard et je l'a remercié pour son travail et lui dire enfin une mesure concrète, enfin une mesure concrète qui allie Sénat proximité et conseils départementaux et c'est ça que nous attendons de la chambre haute et c'est ça je pense que les femmes attendent aussi quelque chose de concret de rapide et d'efficace Moins de 4 mois plus tard, le texte nous revient après avoir recueilli le vote là aussi quasi unanime de l'Assemblée nationale, la lutte contre ces violences notamment faite aux femmes est un combat qui concerne toute la société, c'est un combat universel ce combat me tient particulièrement à coeur comme vous tous mes chers collègues ici présents. En effet je suis engagé pour les victimes comme parlementaire il y a maintenant près de 10 ans, notamment aux côtés de Me Nathalie Tomasini et du juge Édouard Durand que je veux saluer et je sais qu'un certain nombre d'entre vous tente de faire évoluer aussi notre législation. Je pense notamment à notre délégation aux droits des femmes avec sa dynamique présidente Annick Billon que je veux saluer pour son investissement et son énergie pour cette cause. Mais malheureusement ce combat n'avance jamais assez vite. Voilà des années que nous demandons une grande loi sur les violences conjugales et pas d'examiner les choses de façon tronçonner mais voilà plusieurs années que nous devons nous contenter de propositions de lois successives et ce malgré le Grenelle des violences conjugales de 2019. Et comment ne pas évoquer la grande loi du 9 juillet 2010 à laquelle Valérie Létard d'ailleurs et moi-même nous avons participé sur les bancs de l'autre assemblée. Celle de Guy Geoffroy qui a crée notamment l'ordonnance de protection l'expérimentation sur le bracelet électronique, il l'a fait rentrer enfin concrètement dans la loi, c'est la première fois le téléphone grave danger. Ou encore les lois du 28 décembre 2019 et du 30 juillet 2020 qui prévoit, notamment, les dispositions pour améliorer l'accès au logement des victimes de violences conjugales et modifier le régime d'ordonnance de protection prise par le juge des affaires familiales sans oublier les dispositions qui facilite la suspension et le retrait de l'autorité parentale du parent violent mesures que je réclame depuis des années et qui ont été systématiquement systématiquement malheureusement Madame la Ministre rejetée par les gouvernements Hollande et Macron avant d'être intégré. Quelques années plus tard d'ailleurs dans quelques semaines nous aurons à nouveau à examiner un texte à ce sujet je crois Madame la Ministre que ces grandes causes méritent que nous dépassions définitivement de clivages politiques. Il serait temps aussi, rappelons-le, l'analyse des appels du 39 19 révèlent ces dernières années une aggravation des viols conjugaux des menaces de mort et des tentatives de féminicides en 2019 plus de 2100 auteurs de violence en était déjà rendu coupa par le passé aussi. Le texte de notre collègue Valérie Létard crée une aide financière d'urgence aux victimes de violences conjugales, l'aide peut être versée sous forme d'un prêt sans intérêt comme le prévoyait le texte issu du Sénat me mais peut également être un don et il responsabilise aussi le violent conjugal et ça c'est vraiment primordial. Qui devra rembourser à l'issue de toutes les procédures et c'est bien que ce. Qui c'est c'est quand même une avancée aussi considérables qui qui fait en sorte que cette responsabilisation et cette culpabilisation, hé bien elle rentre de façon concrète. Bien sûr, ce texte ne suffira pas à résoudre toutes les failles mais c'est une avancée importante et je veux rappeler qu'un rapport de l'Inspection générale de la justice en 2019 sur les homicides conjugaux âge indique que si 41% avaient alerté les forces de sécurité, 82% des mains courantes à l'époque puisque maintenant c'est différent et des procès-verbaux de renseignement judiciaire n'avait donné lieu à aucune investigation, tandis que 80% des plaines plainte pardon avait déjà abouti à un classement sans suite. C'est pourquoi il est important que nous regardions dans chaque commissariat dans chaque lieu d'accueil comment les choses évoluent et c'est pourquoi nous ne disons pas assez mais avant d'envisager d'autres réformes. Je crois qu'il est nécessaire et vital d'appliquer les lois existantes et de vérifier leur effectivité leur application. Je vais citer un exemple, la loi de 2019 sur les violences conjugales a permis la mise en place d'un comité de pilotage chargé de suivre le déroulement des différentes expérimentations ce comité, dont je suis membre qui devait se réunir. Qui devait réunir de députés et de sénateurs ne s'est réuni que 2 fois en 4 ans. Alors, mes chers collègues. La loi et la justice ont le pouvoir et même la responsabilité de protéger ses victimes. C'est pourquoi bien sûr. J'espère que nous adopterons à l'unanimité cette très belle loi merci beaucoup.

monsieur le Président. Madame la Ministre. Madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. Il y a quelques mois, en octobre dernier, le Sénat a. À l'unanimité la proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes des violences conjugales. Cette initiative sénatoriale constitue à mes yeux un cas d'école. Elle vise à intégrer dans la loi des pratiques qui ont fait leurs preuves sur le terrain, c'est bien sûr le cas du nord et je veux remercier Valérie Létard pour son travail. l'expérimentation menée dans l'arrondissement de Valenciennes et déjà couronné de succès. Si tant est que l'on puisse parler de succès dans la lutte contre les violences conjugales. Dans mon département de la Seine-et-Marne, la CAF a également mis en place. Un système d'aide complémentaire aux victimes de violences conjugales. De toute évidence ce mécanisme d'aide aux victimes fonctionne. Les acteurs de terrain s'en sont emparés. Nous ne pouvons pas l'ignorer. C'est pourquoi je tiens à remercier Valérie Létard pour son initiative qui répond précisément aux problématiques du terrain, les acteurs du du social qui agissent pour la protection des victimes, ont montré leur appétence c'est leur intérêt pour ce type de mécanisme comme lors de la première lecture notre groupe votera en faveur de ce texte afin de permettre la mise en oeuvre rapide. Ce dispositif. Je me réjouis que l'Assemblée. Est également adopter ce texte et que le gouvernement a choisi de le soutenir. Ce soutien est décisif parce qu'il témoigne de la volonté partagée de voir ce dispositif complété toutes les actions déjà mises en place par le gouvernement. L'examen à l'Assemblée a permis de corriger les quelques lacunes du texte que nous n'avons malheureusement pas pu corriger en première lecture, à cause de la, l'article 40 de la Constitution, c'est le cas pour l'intégration des Mutuelle sociale agricole au dispositif qui est désormais acquise. Ce texte met en place des outils nouveaux et je me réjouis qu'il fasse l'objet d'un consensus politique large cependant ce sujet délicat, ne doit pas servir de véhicule législatif pour d'autres combats que celui mené pour la protection des victimes de violences conjugales. C'est pourquoi j'avais déposé un amendement. Que j'ai retiré avant la séance. Ceux d'objet était de modifier à la marge, la rédaction de l'article 1er terre cet article vise à instaurer une loi de programmation pour lutter contre les violences faites aux femmes. Notre groupe est plutôt favorable au principe d'une telle loi de programmation qui permettra de mettre en cohérence les objectifs et les moyens mobilisés à cette fin. Cela nous donnera l'opportunité d'en débattre de façon régulière et sérieuse mais nous regrettons que la rédaction proposée à l'assemblée ne soit pas aussi appropriée que celle du texte initial, en effet, le texte initial, prenez soin de ne pas distinguer entre homme et femme pour s'intéresser à toutes les victimes. Cette modification sémantique est importante car elle introduit un biais idéologique dans ce texte, je crois que notre travail doit rester guidé par le bon sens et la volonté d'aider toutes les victimes de violences conjugales, qu'elles soient des femmes ou des hommes. Même si les deux s'est avéré que l'immense majorité des violences conjugales sont commises par des hommes. Contre des femmes, les violences n'en sont pas moins graves lorsqu'elles ne se sont pas commises contre des femmes je pense là aux hommes qui subissent des violences de la part de leur conjoint tout de leurs conjoints, cela peut arriver. En conclusion, je crois que cette proposition de loi créant tu aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales était essentiel et répond aux préoccupations actuelles de notre société. J'espère que nous pourrons encore améliorer ce texte, même si le plus important est que sa mise en oeuvre sur le terrain, soit la plus rapide possible. C'est ce que les victimes attendent. Merci cher collègue là. Parole est maintenant à madame Mélanie Vogel. Pour le groupe écologiste pour 4 minutes. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, chers collègues. Sous leurs coups sous leurs abus une femme meurt tous les 3 jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables. C'est ce qu'avait constaté Emmanuel Macron le 25 novembre 2017 quand il promettait de faire de l'élimination, l'élimination des violences faites aux femmes la grande cause de son premier quinquennat. Des actes certes mais si peut-on malheureusement suivi cette annonce et quoi qu'on en dise, une chose est claire, l'objectif d'éliminer les violences faites aux femmes n'a pas été atteint, 213.000 femmes sont victimes de violences conjugales en France chaque année 147 féminicides en 2022. C'est 25% de plus qu'en 2021. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est un fait, implacable, les féminicides n'ont pas baissé. Et au contraire ils ont en réalité augmentée. C'est aussi pour cela que les parlementaires ont pris le relais et ce n'est pas rien, je crois, de débattre aujourd'hui d'une proposition de loi et non d'un projet. Je salue donc encore la proposition de loi de Valérie Létard et je veux la remercier encore une fois d'avoir proposé ce texte une étape importante dans le combat contre les violences faites aux femmes par leur conjoint ou ex-conjoint avec mon groupe, je peux vous en assurer, nous soutenons votre proposition et comme en première lecture nous voterons en faveur de ce texte. Ce texte est important parce que il vise à traiter un des grands obstacles à la mise en sécurité des victimes de violences conjugales, qui est la barrière économique. Le revenu des femmes en moins en moyenne inférieur de 22%, celui des hommes. Même si nous sommes plus. Et dans les couples hétérosexuels. L'écart est encore plus grand. Les hommes gagnent en moyenne 47% de plus que leur conjointe et dans cette inégalité se loge le mécanisme de la dépendance, l'absence d'autonomie financière encore plus effrayante lorsque des enfants sont en jeu et donc un déblocage majeur au départ des femmes victimes de violences au delà des inégalités de revenus. Il existe par ailleurs dans ne nombreux cas de violences conjugales, des violences économiques, c'est-à-dire la mise en place d'une stratégie d'emprise financière sur la victime par exemple l'absence d'accès au compte de pouvoir décisionnel financier le contrôle des dépenses et cetera. Et ses mécanismes. Se mettent souvent en place lorsque l'éventualité d'un départ effleure les conjoints violents. Or on sait que nous sommes là autour de la rupture et du départ, au moment de l'annonce de la séparation ou de la survenue de sa crainte chez le conjoint violent au moment le plus dangereux pour la victime de violences car c'est là à ce moment-là qu'elle risque le plus la mort les féministes long collés sur les murs, elle le quitte, il la tue en prévoyant des aides financières pour les femmes victimes de violences conjugales. La proposition de loi vise justement à trouver une réponse à ces situations dramatiques. Dans la première version du texte. la participation financière n'était proposée qu'en terme de près aux femmes victimes de violences. Et pouvait donc constituer une dette à rembourser, dès la première lecture, j'avais souligné avec mon groupe que on ne pouvait pas se limiter à un pré-comme l'ont d'ailleurs fait mes collègues écologistes à l'Assemblée nationale. Je salue donc le fait que, comme nous l'avions en première lecture et grâce à la mobilisation de nos collègues à l'Assemblée à la volonté au soutien de la ministre qui a bien voulu lever le gage est autorisé un certain nombre de d'avancer favorable. Le texte prévoit désormais une aide financière d'urgence aux victimes de violences conjugales qui peut prendre la forme d'un prêt ou d'une prestation non remboursable. Je me félicite aussi que désormais le montant de l'aide puisse être modulée selon selon l'évaluation des besoins de la personne. Et que le remboursement puissent être imputés aux auteurs de violence. Enfin, je rappelle que ce texte ne peut être qu'une première brique car notre horizon politique, ça doit être la diminution des cas de violences eux-mêmes et pour cela, toujours la même chose. Nous demandons que 2 milliards contre les violences de genre du PIB pour protéger 50% de la population. C'est ce que nous continuerons à demander pour la prévention pour la formation pour les mises à l'abri pour que le décompte macabre des féminicides cesse de nous hanter. Je vous remercie. Merci cher collègue là. Parole et maintenant madame Nadège avait pour le groupe RDPI pour 4 minutes. Monsieur le président, madame la rapporteure Madame la Ministre, mes chers collègues. Le texte que nous. Elle mène examinons ce matin en 2ème lecture et que nous nous apprêtons à adopter définitivement en temps créer une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. En tout, 1er lieu je veux ici saluer l'engagement de la vice-présidente du Sénat Valérie Létard. À l'initiative de cette proposition de loi. Mon groupe se prononcera comme il l'a fait en première lecture en faveur de ce dispositif pertinent et déjà expérimenté madame la sénatrice dans votre département. Notre approbation est d'autant plus assuré que le dispositif a répondu à certaines des encres interrogations dont nous avions fait part et sur lesquelles je reviendrai plus tard cette proposition de loi prévoit donc un soutien financier de les conditions d'octroi ont été précisées, ici en octobre dernier rendu accessible rapidement dans un moment d'urgence. Il doit permettre aux victimes en souffrance d'être accompagnées lorsqu'elles prennent cette décision difficile de quitter l'environnement violent. Cette prise de décision dans ma notamment en raison d'une dépendance financière, nous le savons peut être retardé, voire même empêché et cela il faut l'éviter absolument. C'est pourquoi cette nouvelle aide prendra la forme d'un prêt à taux 0 versés en 3 mensualités. Les versements se feront soit par la Caisse d'allocations familiales, soit par les caisses de mutualité sociale agricole dans un délai de principe de 3 à 5 jours ouvrés, après la demande. Le texte prévoit l'application de cette loi dans les départements et régions d'outre-mer nous nous en félicitons. Enfin, nous l'avions souligné préalablement, la notion de près pouvait être source d'insécurité pour les personnes les plus précaires. Les modifications apportées à l'Assemblée nationale ont permis de répondre à notre inquiétude en prévoyant que cette aide pourrait être non remboursable en fonction de la situation financière et sociale et le cas échéant de la présence d'enfants et c'est une belle avancée. Je rappelle ici les chiffres glaçants. Il faut les regarder en face son 22 féminicides au sein du couple ont été recensés en 2021 près de 160.000 plaintes pour violences conjugales enregistrées en 2020 et l'arrêt réalité pourrait être proche du double. Si la règle première en droit civil et pénal et de sortir l'auteur des violences du domicile conjugal et non la victime dans les faits c'est la victime qui va d'abord s'en aller, nous le savons et il faut le prendre en compte cette avance financière doit aussi pour jouer tout son rôle. Aller de Pair avec un accompagnement social et professionnel. Cela est prévu, et elle doit aussi être connue et accessible. C'est pourquoi l'article 2 prévoit que l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit une plainte devra en informer la victime. Il devra également enregistré la demande et la transmettre à la CAF compétentes ainsi qu'au conseil départemental, chef de file de l'action sociale. Il sera important de pouvoir évaluer le fonctionnement de ces le pneu modalités d'accompagnement et cela est également prévue. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera bien évidemment ce texte et je voudrais conclure par le rappel d'une autre information essentielle le 39 19 et le numéro national d'écoute téléphonique et d'orientation à destination des femmes victimes de violence mais aussi de leur entourage et de leurs témoins le 39 19 est anonyme et gratuit 39 19 rappelons-le encore et toujours. Je vous remercie. Merci cher collègue là. Parole est maintenant monsieur Max Brisson. Pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, madame la ministre madame la rapporteure monsieur vice-président de la commission. Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes. Chère Valérie Létard, mes chers collègues. Depuis 2019, le Sénat débattu de plusieurs textes majeurs sur les violences conjugales. Accélération de la délivrance des ordonnances protection renforcement du déploiement des bracelets anti-rapprochement était téléphone grave danger levée du secret médical attribution facilitée de logements d'urgence. Autant de mesures désormais gravé dans la loi et dans la mise en oeuvre parfois trop frileuse a commencé l'accélération de la cadence des travaux du Parlement attestent dans tous les cas du de prise de conscience profonde de l'urgence à agir. Ces diverses mesures ont tenté de compenser quelque peu le retard que nous avons pris sur ce sujet ô combien majeur et quel retard quand on pense que dans notre pays. La première étude statistique sur les violences conjugales. Ne date que de 2006. Cependant, malgré un volontarisme aux politiques récents et des moyens supplémentaires. La croissance du nombre de Willemse conjugal demeure les difficultés inhérentes à leur prise en charge persiste et les crimes violents continuent de briser des vies et des familles. Nous devons continuer les efforts intensifier encore la lutte contre le fléau des violences conjugal. Dans ce contexte, cette proposition de loi instaurant une aide d'urgence une avance sans éthérées ou une aide de mise en place aisée que Valérie Létard a justement voulu universel. est la bienvenue. Une aide pour aider les femmes à quitter une personne violente et à des doit douaniers dans la durée. Mes chers collègues, plus encore que Bienvenue elle sonne comme une évidence dans cette aide est primordiale, primordiale parce qu'elle envoie un message fort, dans un moment particulièrement éprouvant pour la victime. Nous savons s'extraire de l'enfermement que l'on subit au côté d'un compagnon violent est un saut dans l'inconnu. Ce moment-là, celui de la rupture et souvent le plus dangereux c'est là que tout peut basculer vers le drame et c'est précisément pour ces raisons que de nombreuses victimes préfèrent le statu quo aussi insupportable soit-t-il. l'aide universelle d'urgence permettra donc de lever une partie de cet inconnu et de soutenir les victimes dans cet acte de courage primordial aussi parce qu'elle ne répondra pas seulement à des besoins matériels essentiels. Elle donnera le signal d'un soutien de la société à la victime dans une situation de crise elle Camorra la compréhension de leurs difficultés. Elle apportera une réponse aux questions matérielles qui retarde ou pire encore, empêche la victime de violences conjugales de briser l'emprise.

Je salue donc cette avancée majeure qui nous rassemblent pour faire progresser l'aide aux victimes de violences conjugales. Je salue tout particulièrement notre collègue Valérie Létard qui a porté cette proposition de loi issu d'un travail de terrain collectif qui a conduit à imaginer ce système d'avance, indispensable pour que les victimes sortent de la dépendance matérielle que leur impose leur conjoint violent. Au delà du dispositif qui sera créé la. La méthodologie emprunter pour aboutir à l'instauration de cette aide est exemplaire. Elle se fonde sur l'écoute de l'ensemble des acteurs intervenant dans les domaines du médico-social du soutien psychologique de l'aide juridique du logement et de l'insertion professionnelle, la manière dont a été pensé ce dispositif. Nous rappelle qu'à ma Pierre de violences conjugales, seule une approche multi-du dimensionnelle avec notamment les collectivités locales. Les associations, les travailleurs sociaux, les services de gendarmerie, de police, les procureurs de la République et les caisses d'allocations familiales, permet d'aboutir à des dispositifs pertinents. Je souhaite donc qu'à l'aube du chantier majeur qui est celui de la création d'une juridiction spécialité. Que j'appelle de mes voeux regard en particulier tout ce que je peux observer en Espagne voisine, mon département, nous nous souvenons de la pertinence de cette méthode comme d'ailleurs pour tous les autres chantiers cas recensés fort justement il y a un instant, Laurence au signal que nous nous souvenons de l'urgence d'agir, mais aussi de créer consensus pour intensifier encore la lutte menée contre les violences conduit de Galles qui nécessite d'encore mieux coordonner les acteurs et de supprimer ces terribles trous dans la raquette dans laquelle malheureusement s'engouffrent encore trop souvent les auteurs. Dans l'attente. Madame la Ministre d'une grande loi de lutte contre les violences conjugales, le groupe Les Républicains votera bien entendu conforme. Cette proposition de loi attendu et utile. Merci cher Valérie d'État. Qui est contre. Chers collègues, en dehors des articles de bis trois qui sont supprimés, est-ce que je peux considérer en les appelant naturellement. Que le vote est identique sur tous les articles. Oui donc article 1er bis article 1er article de de terre de quater de qu'inquiète. Sont adoptés et je mais aux voix l'ensemble du texte de la proposition de loi qui est pour.

Chavanel au nom de la prendre. La commission des social vous remercier vous féliciter pour pour les travaux mais d'une façon générale. Je voulais remercier l'ensemble des sénateurs pour leur mobilisation sur cette grande cause qui nous anime tous et donc c'est l'occasion pour à la fois de remercier et féliciter et de porter un excusez-moi les sénatrices et les sénateurs. C'est bien la remarque est importante. Excusez-moi et je voulais en profiter notamment pour porter un message auprès de Madame la Ministre pour vous dire que d'une façon générale cette unanimité porter ici dans l'hémicycle montre combien le sujet nous anime tous et je crois qu'il est vraiment important et urgent que nous ayons et les sénatrices et les sénateurs. L'occasion de pouvoir vous accompagner dans un texte global sur les violences véto femme c'est une volonté à la fois de la commission mais d'une façon générale du Sénat et vous aurez ici des partenaires dans l'unanimité dès lors que nous aurons tous la capacité de nous mobiliser quelques sonore en c'est un message que je voulais porter. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Monsieur le président, mesdames les sénatrice mesdames les sénateurs. Moi aussi je suis ému. De l'adoption de cette proposition de loi à l'unanimité. Alors, bien sûr. Merci cher Valérie Létard pour cette proposition. Merci pour pour la qualité de nos échanges aussi. Merci à Madame la rapporteure chers Jocelyne Guidez pour pour tout le travail effectué. Je suis heureux aussi que nous ayons pu ajouter donc la possibilité du don un. Sous pour la forme de cette aide universelle d'urgence à laquelle nous nous tenons vraiment très fermement. Et puis nous allons maintenant nous attaquer à l'élaboration du décret

le travail constant et toujours constructif que nous menons avec la la délégation aux droits des femmes et notamment sa sa présidente cher Annick Billon et puis bien sûr le travail. Continue. Laurence Rossignol Marc Marc Max Brisson et vous savez combien pour moi cette notion de justice spécialisée est fondamental je maintiendrai toujours que ces violences ne sont pas des infractions comme les autres et qu'elle nécessite un traitement et une prise en charge spécifique. Nous, nous allons bientôt. Pouvoir recevoir le le rapport justement effectué par les 2 parlementaires que sont donc la sénatrice Dominique V. rien et la députée Émilie Chandler sur ce sujet et vous pouvez compter sur moi je sais aussi que je peux compter sur sur vous. Je pense que nous avons vraiment un message unique aujourd'hui c'est que face à ces violences. Eh bien, seule l'union fait la force. Voilà, merci à vous toutes et tous. Merci, madame la Ministre. Changement d'équipe si je puis me permettre.

me permettre. Du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports et de l'agriculture. La parole est immédiatement madame la présidente. Pascale Gruny rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire pour cinq minutes. Monsieur Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. La commission mixte paritaire réunie le 9 février dernier est parvenu à un accord sur le projet de loi Dadu qui adapte notre législation droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports et de l'agriculture. Je salue la rapporteure de la CMP pour l'Assemblée nationale, ainsi que l'ensemble des rapporteurs des 5 commissions qui se sont saisis sur ce texte en première lecture. Leurs travaux ont permis de compléter ce projet de loi et de trouver un accord entre nos deux chambres. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des dispositions du texte dont nous avons discuté en première lecture et qui pour nombre d'entre elles n'ont été modifiés que très marginalement, par l'Assemblée nationale. J'évoquerai les principales modifications adoptées par la commission mixte paritaire. En matière de handicap. La CMP a intégré l'apport du Sénat, visant à ce que le renouvellement des terminaux en libre-service pour les rendre accessibles aux personnes handicapées soient effectuées en s'assurant d'une répartition territorial équilibré. L'égalité d'accès des personnes atteintes d'un handicap au service de la vie courante comporte une dimension territoriale qui devait être prises en compte. Concernant la santé la CMP n'a apporté qu'une précision sur les catégories de personnes et de services autorisés à délivrer des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spécial. Dans le Champ de l'économie, nous avons apporté plusieurs modifications à l'article 5 bis hein qui porte sur l'encadrement des prestataires de services sur actifs numériques. Un mécanisme d'enregistrement renforcée de ses prestataires auprès de l'Autorité des marchés financiers. L'AMF a été retenue qui exigera des prestataires qui dispose d'un système d'enfants informatique résiliant et sécurisé. Pour que tous les nouveaux entrants sur le marché dispose d'un enregistrement renforcée au 1er janvier 2024. La CMP a fixé au 1er juillet 2023, le délai limite pour le dépôt des dossiers des prestataires souhaitant demander un enregistrement simple. En matière de transport, la CMP encadrer la possibilité donnée à l'Autorité de régulation des transports de procéder à des collectes automatisé de données publiquement accessibles sur des services numériques de mobilité. Un avis de la CNIL sera rendu sur le décret d'application du dispositif et ses collègues seront mises en oeuvre de manière proportionnée et strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de cette autorité. Enfin concernant l'agriculture, la CMP a précisé les conditions d'attribution des aides à l'installation des agriculteurs versée par les régions. Les jeunes agriculteurs et nouveaux agriculteurs pourront bénéficier de ces aides, à condition à condition de justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'un digne d'un niveau de diplôme ou d'expérience professionnelle. Préalablement à leur installation par dérogation ce niveau pourra être atteint progressivement par le candidat au cours de l'installation. Telles sont les principales modifications intervenues en commission mixte paritaire. Je vous invite donc, mes chers collègues à adopter le texte résultant de ces travaux et je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est maintenant à Madame Olivia Grégoire Ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Vous avez la parole. Madame la ministre. Madame la rapporteure. Messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis ce matin. Afin que la chambre haute puisse adopter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi. Portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports mais aussi de l'agriculture. Au nom du gouvernement. Je tiens d'abord à vous remercier d'être parvenu avec les députés à cet accord important, vous le savez. Ce projet de loi a pour objet de transposer de mettre en oeuvre un certain nombre de directives et de règlements que l'Union européenne a adopté ces 3 dernières années. Il procède également à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendue nécessaire. Le texte à bord d'un nombre très variées, comme a dit la madame la rapporteure sur des sujets sur lesquels je ne reviendrai pas techniquement de manière exhaustive. Vous avez déjà eu tout loisir d'en débattre. Le projet de loi va pêle-mêle permettent la mise en oeuvre résume pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués DLT qui entrera en application dès le mois de mars pour une durée de 3 ans. La France s'est battue pour obtenir un régime pilote ambitieux qui permette de conduire des expérimentations à taille industrielle sur les usages de la bloque chaînes. Et le gouvernement se réjouit aussi de pouvoir disposer d'un régime créant une zone d'expérimentation. Pour lui. Utilisation de la technologie Blockchain dans le domaine des instruments financiers. Déterminant pour rester dans la course des innovations financières à l'échelle mondiale, la place de Paris d'ailleurs pourrait aujourd'hui devenir la place de la mise en oeuvre du régime pilote et en tirer un Avantage comparatif substantielle. Je m'arrête également un instant sur l'article 5 bis qui a été introduit dans nos débats par le Sénat. Et qui traite de l'évolution des règles qui s'appliquent aux acteurs souhaitant s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers comme prestataire de services sur les actifs numériques. Le gouvernement prend acte à regret que l'accord trouvé entre députés et sénateurs soient plus dur notamment en terme de calendrier que la position du gouvernement et des régulateurs. Je ne peux m'empêcher d'évoquer aussi l'article 8 portant transposant la directive. SRD. Sur les rapports extra-financiers. Dont je sais qu'il a fait fort débat ici. Pour des raisons qui honore le Parlement. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de longuement débattre dans ce même hémicycle il y a quelques semaines avec vous sur les opportunités que revêt cette évolution en matière de performance extra-financière de nos entreprises dans le cadre d'un débat très intéressant. Sur la responsabilité sociale de nos entreprises, le gouvernement et votre serviteur. En premier lieu et vraiment satisfait que la CMP maintenu cet article et continuera de travailler en transparence avec les parlementaires qui le souhaiteront, sur les suites de cette habilitation importante je veux aussi mentionné l'article 12 qui a quasi intégralement évoluer d'une habilitation vers une écriture de la transposition de la directive accessibilité des produits et des services pendant la navette parlementaire comme le gouvernement s'y était engagé. C'est un pas important pour nos concitoyens en situation de handicap et donc pour toute notre société. Sur ce sujet. Qui me tient à coeur, on a tous nos raisons, et nos sujets qui nous tiennent à coeur en politique sur ce sujet qui me tient profondément à coeur nous accusons un retard collectif qui n'est pas acceptable et je veux saluer sincèrement le travail technique, exigeant que ces transpositions à impliquer Le texte contient par ailleurs de nombreuses dispositions relatives aux prérogatives des ministères sociaux je pense à l'article 14 qui portent des mesures concernant le congé parental d'éducation. Le congé de paternité. Le congé de solidarité familiale et de proche aidant et qui a pu évoluer dans le cas de la navette parlementaire, je sais. Et je vous en remercie. Madame la rapporteure que vous êtes très engagé sur cet article et je veux aussi la très sincèrement saluer le travail du Sénat. L'article 23, quant à lui permet de ratifier des ordonnances désignant l'autorité administrative chargée de prononcer des sanctions financières dans le cas de la surveillance des du marché des dispositifs médicaux des dispositifs médicaux de diagnostic in utero et de leur as accessoires là aussi. Là encore, le Sénat a travaillé ardemment à l'amélioration des outils de lutte contre les risques de rupture de dispositifs médicaux et à la possibilité de publier les éventuelles sanctions financières prononcées par l'autorité par l'autorité administrative en la matière le gouvernement salue ce travail enfin le projet de loi comporte un certain nombre de dispositions relatives au secteur des transports dont je sais qu'elles ont suscité une mobilisation particulière de la part des sénateurs ainsi que de nécessaires mesures d'adaptation du code rural et de la pêche maritime à la mise en oeuvre de la programmation 2023 2023 27 de la Pac dont vous savez qu'elle est un outil vital pour nos agriculteurs, vous l'avez compris, en un mot le gouvernement vous remercie mesdames, messieurs les sénateurs pour le travail accompli sur les différentes dispositions de ce texte, un texte technique mais aussi très riche, variée et je sais que nous partageons l'ambition que ces mesures se concrétise rapidement pour le quotidien de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci madame la ministre. Et merci pour vos remerciements à la Haute Assemblée. Je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat étant appelés à se prononcer avant l'assemblée nationale il statue sur les éventuels amendements puis par un seul vote sur l'ensemble du texte. En conséquence, nous passons à la présentation puis au vote de l'amendement du gouvernement avant d'en venir aux explications de vote, des groupes. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Cet amendement est un amendement de coordination pour adaptation aux articles ultramarins. Il s'agit donc d'un amendement de cohérence dont je ne doute pas qu'il l'emportera votre adhésion. Je vous remercie. Il y avait de la commission, madame la présidente. c'est un avis favorable bien entendu puisque c'est la cohérence et que pour. Nos amis ultramarins c'est c'est important. Et nous l'avons pas vu en commission. Mais bien sûr ce c'est un avis très favorable. dans le jeu mais au voilà l'amendement 5 bis du gouvernement avec avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Nous passons aux explications de vote, des groupes à raison d'un orateur par groupe. Monsieur Pascal Savoldelli pour le groupe CRCE pour cinq minutes.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues. Ce projet de loi vise à conformer notre droit au droit. De l'Union européenne. Et là on assiste à un catalogue de régression droit financier de dispositions contraires à l'intérêt général et de recul en matière de droits sociaux Des avancées adopté au Sénat mais curieusement non défendu en commission mixte paritaire on atterrit sur un texte sans amélioration majeure pour lequel nous voterons contre. Et plus d'eau plutôt 2 fois qu'une. Je souhaite alerter sur 3 aspects le 1er un ajout du sénateur Hervé Maurey qui souhaitaient soumettre à agrément préalable de l'autorité des marchés financiers tout acteur voulant exercer la profession de prestataires de services sur actifs numériques. Que n'avait-il pas osé faire en demandant de rendre obligatoire la délivrance d'un accord facultatif. Aussi bien les échanges en CMP. Que les réactions des acteurs du marché de leurs représentants et l'hostilité du gouvernement. Nous on a paru complètement déconnectée de l'intérêt d'agir. Je m'excuse mais il faut cesser d'opposer, innovation technologique et régulation. Prenons un exemple, la société biquette elle proposer un service d'achat d'un coupon chez son buraliste en espèces pour ensuite recevoir des bitcoins. L'autorité de contrôle prudentiel met en avant je cite des débits au portefeuille des clients sans leur consentement ou encore je cite des défaillances sérieuses du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Sans parler d'un vol de 300.000 euros. L'enquête est en cours. En résulte une radiation par l'AMF le 28 septembre. Pourquoi cet exemple Bakiev c'était simplement enregistrer. Elle ne disposait pas du fameux agrément et donc sans contrôle préalable exigeant de l'AMF. Le compromis trouvé en CMP et moins 10 ans mais permettra à terme dans l'attente de la directive européenne. Mika de limiter les dérives de secteurs un secteur aussi innovant technologiquement que frauduleusement 2ème aspect l'article 8 supprimé par le Sénat rétablit à l'Assemblée nationale sur la possibilité de transposer par Ordonnance la directive sur la durabilité des entreprises. Il se trouve que la rédaction de cette directive n'est pas terminée. Et nous attendons toujours les actes délégués entre l'article 7 fondamentales sur la transparence sur le revenu des entreprises, pays par pays et celui-ci, cela fait beaucoup et beaucoup trop d'habilitation, concrètement pour l'article 7 on transpose trop tard et pour l'article 8 on transpose trop tôt. Il y a un juste milieu. C'est un projet de loi spécifique en dur dans la loi, pas une ordonnance en catimini d'ailleurs le ministre Jean-Noël Barrot ne disait pas autre chose, je le cite, il disait aurait-il mieux valu un texte en dur, peut être. Si la France est en avance sur les obligations déclaratives en matière de performance extra-, financière, sociale et environnementale. Le rapport du Sénat sur le texte rappelle à juste titre je cite le manque de données fiables comparable exploitable facilement pour permettent de comparer les actions menées par les différentes entreprises. C'est l'objectif de la directive, c'est également l'objectif d'une proposition de loi de notre groupe. Oui, nous souhaitons l'abaissement du seuil de publications d'entreprises de plus de 50 salariés et non pas comme le prévoit la directive seulement à celles de 250 salariés et à terme aux PME cotées en bourse. Dans notre groupe, nous considérons que ces informations sont une mine d'or indispensable pour conduire des politiques publiques, la mise en place d'outils fiscaux le pilotage d'aides publiques aux entreprises. Il s'agit pas simplement de sanctionner des entreprises sur la base de leurs déclarations. L'information des citoyens est crucial pour conditionner quand même chaque année 160 milliards d'aides publiques aux entreprises. Les entreprises de plus de 50 salariés ne peuvent pas même de façon agrégé rivaliser et là j'y vais avec BNP Paribas, la Société générale, le Crédit Agricole ou Total. Qui ont une empreinte carbone d'ailleurs supérieure aux éditions de la France. Mais nous savons désormais que nous ne contraindrons pas le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degrés. Les entreprises doivent intégrer plus fortement la réduction des émissions dans leur modèle économique 3ème aspect c'est l'article 11 qui permet à une entreprise. Alors là ça vaut le coup quand même de contourner des décisions prononcées par le juge judiciaire. C'est-à-dire que condamnés pour des infractions pénales des entreprises que je nomme délinquante n'auront qu'à prouver leur bonne foi. Pour bénéficier de nos marchés publics et de l'argent public alors que et je parle avec sérieux. On parle de faits graves. Blanchiment actes de terrorisme traite des humains, fraude fiscale et la liste est longue. Aujourd'hui, en droit français, une entreprise doit attendre 5 années après sa condamnation pour l'un des faits que je viens de mentionner pour recouvrer le droit de soumissionner à un marché public lorsque le droit de l'Union européenne à ce point vicié que la France avait résisté au moment de sa transposition. Le Conseil d'État a interprété le droit, chacun est dans son rôle mais le Parlement doit se dresser. Lorsqu'une disposition est manifestement contraire aux droits humains aux principes et aux valeurs constitutionnelles du préambule de la Constitution de 46 et 58, le Parlement en responsabilité en autonomie doit s'interposer. Merci. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Madame Jocelyne Guidez pour le groupe Union centriste pour cinq minutes.

Monsieur le Président Madame la Ministre monsieur le président de la commission, madame la rapporteure chers collègues nous examinons aujourd'hui. Conclusion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de. L'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports et de l'agriculture. Je salue le travail des rapporteurs et en particulier de Madame, Laurence. Ce qui Christol et notre collègue Pascale Gruny qui ont contribué au bon aboutissement de cette CMP. Je regrette qu'aucun des 31 articles restant en discussion n'a été adopté dans la rédaction du Sénat mais outre des rapprochements concernant des modifications rédactionnelles. Je note que la position du Sénat et en particulier de notre collègue Hervé Maurey a été retenu, premièrement pour les dispositions relatives au domaine de l'économie. La CMP a trouvé un accord privilégiant le renforcement de l'encadrement des prestataires de services sur actifs numériques, c'est-à-dire les cryptoactifs, telles que le bitcoin notamment pour répondre aux risques cyber particulièrement élevé dans le secteur des actifs numériques. Le texte initial d'intégrer aucune mesure en la matière. De même, sur proposition de la commission des finances. Le dispositif sera pleinement opérationnel dès le 1er janvier 2024. Plus globalement, c'est un cas de plus favorable aux épargnants sans entraver l'innovation financière l'approche du Sénat qui a adopté en première lecture un renforcement de la régulation de ces acteurs. Contre Contre l'avis du gouvernement et donc validé cette mesure s'impose, compte tenu des graves dérives dans ce secteur, révélé par une succession de. Intervenues ces derniers mois et notamment la chute de la société MTX qui pourrait avoir lésé plus de un million d'investisseurs. L'Assemblée nationale avait adopté en première lecture un dispositif moins protecteur pour les épargnants que celui proposé par le Sénat. De plus, le Sénat avait voté la suppression de l'article 8 et de son habilitation visant à transposer la directive relative à la publication d'informations de durabilité des entreprises. Nous nous félicitons d'avoir été entendus concernant le recevra du Champ de l'habilitation proposé là proposé là encore par la commission des finances pour sauver une transposition dont les marges de manoeuvre sont réduites. Enfin la CMP a trouvé un point d'équilibre. Quant à la directive sur l'accessibilité des produits et services. Celle-ci sera finalement directement transposer dans notre droit, afin de mieux coller au calendrier de ses obligations. L'accord retient d'ailleurs les dimensions physiques et territoriale de cette accessibilité que le Sénat a tenu à mettre en avant en garantissant que le renouvellement des terminaux en libre-service assure une répartition territoriale équilibrée en vue de leur accessibilité en particulier aux personnes handicapées. Deuxièmement, concernant les dispositions relatives à la santé. L'article 20 sur les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spécial a également fait l'objet d'un consensus bienvenue qui respecte à la fois l'intérêt des patients et des pharmacies en reprenant l'objectif de sécurisation porté par notre assemblée la CMP valide le principe de renvoi. Quant à la loi qu'au pouvoir réglementaire, le soin de constituer la liste des personnes autorisées à délivrer ces denrées la voie réglementaire ne pourra toutefois intervenir que si elle garantit le contrôle médical telle qu'exigée par le droit communautaire en vigueur. Troisièmement pour que pour ce qui est de, des transports, le Sénat a également été entendu dans sa volonté de préciser et encadrer davantage le dispositif de collecte d'automatisée par l'Autorité de régulation des transports des données publiquement accessibles sur des services numériques de mobilité. Cette collecte étant rendues nécessaires par le volume de ces données ainsi que le nombre d'acteurs concernés qui ne permettent pas à l'autorité de mener à bien les missions qui lui ont été confiées dans le cas de la loi d'orientation des mobilités quatrièmement sur le volet agricole de ce projet de loi, l'article 30 entérine. La régionalisation des aides à l'installation des jeunes agriculteurs. C'est effectivement un gage à la fois de flexibilité et d'adaptation au terrain la CMP n'a pas. N'a par ailleurs suivi notre opposition qui consistait à inviter les régions à réaliser un bilan annuel de leur action en tant qu'autorité de gestion des aides à l'installation. Enfin, l'accord entérine rédactions de compromis sur les conditions minimales nécessaires au bénéfice des aides à l'installation. Vous ne vous l'aurez compris, chers collègues, nous voterons en faveur de ses conclusions. Je vous remercie. Merci cher collègue là. Parole et maintenant Monsieur Henri Cabanel pour le groupe RDSE pour cinq minutes.

Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. Marronnier de l'éventail parlementaire ces projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne n'en reste pas moins nécessaire porteur de réelles avancées. Quand bien même leur apparente complexité et technicité. En première lecture, le groupe RDSE attentive à l'expression législative de la solidarité, ainsi qu'à la protection de nos concitoyens français et européens, avait insisté sur la nécessité de rendre plus efficient. Et efficace. Notre société en matière d'inclusivité. Nous partageons les inquiétudes de la commission des affaires sociales du Sénat, qui a estimé que l'enjeu quant à l'amélioration de l'accessibilité d'un certain nombres de produits et services liés aux usages numériques résider davantage dans le calendrier de mise en oeuvre de ces obligations par les opérateurs économiques que dalle, l'adoption et la promulgation de ces nouvelles règles Anne droit interne nous rappelions également au regard des retards constatés dans l'application de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées que le gouvernement devra être volontaire. Quant à la nécessité de prévoir un régime d'incitations voire de sanction de nature à accompagner les opérateurs économiques dans le déploiement des évolutions techniques nécessaires à l'accessibilité des produits et services, notamment en zone rurale. Autant d'inquiétudes auxquelles nos 2 assemblées et la, la commission mixte paritaire ont permis de répondre. Le groupe RDSE se réjouit en effet que les l'effort collectif hein. Vers une inclusivité toujours plus subi que de notre société soit matérialisée par une transposition directe de notre droit et non plus par ordonnance de la directive du 17 avril 2019 relatives aux exigences en matière d'accès d'accessibilité applicable aux produits et services. Cette initiative permettra notamment de respecter le calendrier de mise en oeuvre de ces nouvelles obligations. Et si la mise en confort qui a en conformité des produits et services intervient interviendra dans les les les cours néanmoins acceptable pour les opérateurs et sera soumise à un régime renforcé de contrôle et de sanctions. Par ailleurs, le groupe RDSE tenait à saluer le maintiennent dans le texte après ajout au Sénat de la garantie de la dimension territoriale de l'égalité d'accès des personnes atteintes d'un handicap par ces produits de la vie courante assure assurant ainsi une répartition territoriale équilibrée. D'autre part en matière de transport. Notre groupe se félicite de la transposition de la directive Eurovignette relative à la taxation des véhicules lourds. Empruntant certaines infrastructures routières afin d'intégrer de nouvelles règles de modulation et de majoration des péages applicable à ces véhicules notamment en fonction des émissions de CO2. Je rappelle que le Sénat avait adopté plusieurs demain visant à relever l'ambition du texte en faveur de la transition écologique et accompagner les transporteurs dans le verdissement de leur flotte en permettant notamment d'exonérer de redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique. Les véhicules les moins polluants. Sujet fondamental puisque les autoroutes françaises sont responsables de 7% des émissions de gaz à effet de serre. Du pays, dont 54% de ces émissions provenant des poids lourds jette mesure fait écho à la volonté de notre groupe d'accompagner plus concrètement et rapidement les professionnels du secteur face aux difficultés économiques et structurelles qui rencontrent. Le verdissement de leur flotte et leur adaptation notamment aux nouvelles normes imposées à l'échelle nationale pour les zones à faibles émissions mobilité. Rappelons que le verdissement de la flotte de poids lourds effréné par de multiples facteurs loft industriel de véhicules électriques ou hybrides est encore trop réduite et trop coûteuses sur les segments des véhicules les plus lourds et il y a besoin d'une autonomie élevée. Autant de raisons ralentissent à la transition de ce parc vers des véhicules à basse consommation. Ainsi, si l'homme peut lever les incertitudes technologiques et énergétiques le vont au moins les incertitudes politiques et juridiques, la transposition de la directive Eurovignette. Dans ce cadre et constitue une évolution opportune à l'adaptation de notre société à celle de demain. N'oublions pas que cette démarche doit être incitatives aux évolutions marquées par l'accident l'acceptabilité et la justice sociale et non pas se transformer un ambassadeur d'une écologie punitive. Ne pouvant commenter les articles et notamment pour la première fois ceux liés à l'agriculture. Le groupe RDSE tenait à mettre l'accent sur ces 2 avancées législatives pour une société plus inclusive et efficiente à certaines de ces âges qui nous sont contemporains. Vous l'aurez compris, notre groupe sera favorable pour ce texte. Je vous remercie. Cher collègue, la parole est maintenant monsieur Max Brisson. Pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre Madame la rapporteure, mes chers collègues. Ce projet de loi rassemble des dispositions très diverses et leur seul point commun réside dans l'urgence à les intégrer dans notre droit. Dans ce contexte, je tiens à saluer le travail des rapporteurs contraint d'examiner les aspects techniques du projet de loi en un temps très limité. La commission des affaires sociales et ainsi soutenu les avancées concrètes du projet de loi visant les personnes en situation de handicap. Les salariés ou encore les patients concernant l'accessibilité des personnes handicapées. La CMP a notamment retenu le souhait du Sénat de 41 répartis second territorial équilibré des terminaux en libre-service tels que les distributeurs automatiques de billets ou de titre de transport en droit du travail ont été ajoutés les périodes de congés de paternité parmi les périodes de congés assimilée à une présence d'entreprises, ce qui permettra de compter ce congé pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés comme nous avions déjà pour l'intéressement. L'année dernière. La question du contrôle des denrées alimentaires destinées à défaire médicale spécial a fait l'objet de débats nourris les exigences à respecter, ont pu être renforcée. Concernant l'approvisionnement en dispositifs médicaux. Je salue la mesure proposée par notre rapporteur Pascale Gruny contraignant les opérateurs à prendre les mesures nécessaires lorsqu'il constate un risque de pénurie ou informés en un mot, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ou des produits de santé qui prendra toutes mesures utiles ces ruptures ont en effet tendance à s'accroître, sans que quiconque ne dispose d'une information claire à ce sujet et sans qu'aucun mécanisme qui était prévu pour les prévenir. À la différence des médicaments alors que ces ruptures peuvent avoir des conséquences graves pour les patients. La commission des affaires économiques à l'initiative de son rapporteur Laurent Duplomb assez quant à elle, intéressée aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs en imposant notamment un bilan annuel des installations par chaque région le renouvellement des générations est en effet devenu un enjeu majeur de notre stratégie agricole sachant que 43% des agriculteurs ont atteint l'âge de départ à la retraite d'ici 2030, à raison d'une position divergente de l'Assemblée concernant notre souhait de formation du jeune agriculteur. La commission mixte paritaire à trouver une solution de compromis permettant régions par dérogation d'attribuer des aides au cas par cas à des personnes qui ont atteint le niveau nécessaire en cours d'installation. La commission des finances. Elle a poursuivi le travail d'harmonisation des dispositions applicables aux mutuelles aux institutions de prévoyance et aux sociétés d'assurances. D'autre part un article, introduit par son rapporteur rêver Maurer est venu traiter la question du régime applicable au prestataire de service sera kif numérique le Sénat souhaitait imposer aux acteurs l'obligation de demander l'agrément aujourd'hui facultatives délivrées par l'Autorité des marchés financiers plutôt que gréement. Les députés ont opté pour une enregistrement. Ils ont repris les exigences que nous avions mentionné ce dispositif devrait entrer en vigueur rapidement au 1er janvier 2014 comme le souhaitait le Sénat, la commission des lois à elle utilement compléter l'habilitation à transposer la directive de 2017 concernant les transformations fusions et scissions transfrontalière son rapporteur Didier Marie à encadrer les choix de transposition du gouvernement est contraint celui-ci à agir d'ici 3 mois au lieu de 6. Enfin je voudrais vraie parmi les sujets de la commission du développement durable. Son traitement de la directive Eurovignette permettant notamment la mise en oeuvre d'exonérations ou de réduction des péages au bénéfice des véhicules les moins polluants. À l'initiative du rapporteur Cyril va le Sénat par ailleurs modifié le texte concernant la mise en oeuvre du règlement européen sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Nous avons élargi la protection des voyageurs notamment en obligeant les entreprises ferroviaires. Ainsi que les gestionnaires de gare à indemniser les personnes handicapées ou à mobilité réduite en cas de perdre autant moi je monte leur dispositif d'assistance. Ainsi, malgré leur caractère extrêmement technique, les dispositions du projet de loi auront des conséquences très concrètes pour nos concitoyens le présent texte étant consensuels répondant aux exigences fixées par le droit de l'Union européenne, le groupe Les Républicains votera ce texte, je vous remercie, je vous quelques minutes. Votre président, une minute, une minute. Merci ciao. La parole est maintenant Madame, Colette Mélot pour le groupe les indépendants pour cinq minutes.

Monsieur le Président Madame la Ministre. Madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission. Des affaires sociales. Mes chers collègues. Ce projet de loi portant diverses dispositions d'de dettes. D'adaptation au droit de l'Union européenne a été adopté rapidement d'chacune des assemblées avec un travail rigoureux. C'est ainsi, sans surprise, que nous sommes parvenus en tout juste 2 mois à une CMP conclusive. Il n'en demeure pas moins que ce texte reste très technique et les sujets très variés. Je salue le travail effectué par nos rapporteurs ainsi que par l'ensemble des sénateurs à la fois en commission des affaires sociales et un hémicycle. Lors de la première lecture du texte. Je me suis attaché principalement au volet concernant les affaires sociales notre commission étant saisie sur le fond mais je me félicite de voir que les autres sujets concernant l'économie, le travail, les transports et l'agriculture ait été traité avec la même efficacité. Ces domaines sont essentiels au niveau européen, tout comme au niveau français. Me notre droit en conformité, c'est aussi faire ruisseler le choix les choix positif que nous avons pris à 27 afin d'impacter de la meilleure des façons la vie des citoyens européens. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, de le démontrer, grâce à un rapport sur les fonds européens, l'Union européenne fait partie de notre quotidien et c'est une ah ne chance. Sont là. Pour revenir au sujet, sur lesquels j'avais choisi de m'attarder en décembre dernier et qui relèvent du secteur de la santé du travail. Je suis satisfaite de constater que le texte reste équilibré concernant l'article 14 qui se penche principalement sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et et dans le Sénat a effectué un travail qui a été préservée à l'Assemblée nationale et au et j'insiste à nouveau sur les adaptations apportées en direction des proches aidants, et je tiens à saluer une nouvelle fois leur dévouement à chaque instant. Les dispositifs médicaux et les mesures qui les concernent dans l'article 23, me paraissent également aller dans le bon sens. Le texte garde la volonté principal de l'anticipation particulièrement concernant les problèmes d'approvisionnement des dispositifs médicaux. Cette question est particulièrement crucial au sein de l'Union européenne et pour la France. C'est une question de souveraineté. Plus largement, l'Union européenne ne cesse d'accroître sa place dans notre quotidien. Les décisions qui sont prises depuis l'arrivée de la nouvelle Commission européenne nous impacte directement. Elle cherche à mettre en musique la feuille de route que nous nous sommes donnés collectivement concernant de transition à la fois écologique et numérique. Le dernier conseil européen extraordinaire qui a eu lieu en jeudi dernier est revenu sur la compétitivité et la politique industrielle de l'union de sujets cruciaux pour l'avenir des Européens et notre indépendance dans un monde aux enjeux multiples, une nouvelle de feuille de route est tracée. Des décisions sont prises et des directives et règlements négociés et adoptés in fine ce sera là encore le temps de nouvelles de nouveau projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne sur les domaines toujours aussi divers. J'ai alerté sur la subsidiarité notre vigilance, nous devrons poursuivre nos travaux nous parlementaires nationaux avant un rôle clé pour une application équilibrée de ce principe. J'ai aussi rappelé que pour notre groupe, la surtransposition n'était pas une option, ni même les erreurs de transposition je sais l'engagement de ce gouvernement sur ces 2 points clés. Le texte de ce projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, issu de la CM MP nous semble répondre aux objectifs fixés. Vous l'avez compris le groupe les indépendants votera donc en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Jacques Fernique. Pour le groupe écologiste pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre chers collègues on a voté donc en première lecture il y a tout juste 2 mois en faveur de ce projet de loi de transposition du droit communautaire. Un texte. Hétéroclite qui a mobilisé nombre de commissions et de rapporteurs autant dire pas facile pour chacun d'entre nous dans les délais très restreint que nous avions d'en avoir une maîtrise globale de façon à accomplir notre travail perte parlementaire en connaissance de cause. Après les modifications apportées par nos collègues de l'Assemblée et les ajustements en commission mixte paritaire. Mon groupe estime que son vote positif d'il y a 2 mois peut être réitéré bien entendu, on aurait pu aller plus loin. Mon groupe regrette que ces transpositions soit parfois trop peu ambitieuse. Les directives règlements dont il est question aurait mérité une volonté plus forte afin d'assurer une adaptation optimale dans notre droit. Car si ce texte très disparates et d'une grande technicité. Il va tout de même avoir ça vient d'être rappelé des effets concrets pour les Françaises et Français dans des domaines aussi variés que le droit au travail pour les congés de paternité l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, la santé, les transports, l'agriculture ou encore les publications en matière de durabilité par les entreprises. Je regrette que ce texte ne couvre pas les évolutions nécessaires dans 2 domaines sur lesquels je concentrerai mon propos sur les affaires sociales. Certes, notre groupe salut certaines avancées. Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et proches aidants un renforcement de la coopération entre pays européens en matière de services d'aide sociale à l'enfance des exigences d'accessibilité à certains produits et services en ligne pour les personnes en situation de handicap mais nous regrettons que cela ne s'inscrivent pas dans une stratégie nationale sur l'accessibilité qui serait vraiment nécessaire, c'était la demande du Collectif handicap qui avait regretté de ne pas avoir été associés aux travaux de transposition de cette directive. Il a été en partie entendus avec l'intégration d'un de ces amendements porté entre autres par notre groupe si ce texte, je l'ai dit comprend des avancées intéressantes quant au congé de paternité. D'autres groupes pensent qu'il faut aller plus loin, à l'instar des espagnols. Pourquoi pas cette semaine non transférable pour chacun des 2 parents rémunéré à 100%. Sur les transports. Cette adaptation de la directive Eurovignette actualisées et le moment, je crois, pour prendre enfin conscience pleinement conscience de la situation atypique en Europe d'une France qui n'a que ces péages autoroutiers alimentant les entreprises concessionnaires leur taux de rentabilité très élevée et leurs actionnaires. La France, on le sait, ayant renoncé à une redevance pollueur payeur et à ces portiques sur son réseau principal. C'est pourtant ce que pratique l'essentiel de nos voisins européens. L'adaptation de la directive Eurovignette se borne donc à impacter en service plutôt minimum les seuls péages des hypothétique future concession autoroutière minimum puisqu'on reporte à plus tard les redevances facultative congestion pollution sonore et atmosphérique. Puisqu'on épargne aussi les grands véhicules et utilitaires légers concessions hypothétique puisque le choix du futur modèle d'exploitation des réseaux dont les concessions se termineront d'ici 8 à 13 ans n'est bien sûr pas encore fait. Mise en régie, poursuite des concessions avec quelle durée. Autre forme de partenariat public-privé. Quel que soit le choix, les péages actuels seront remis en question et le président du conseil d'orientation des infrastructures de transport nous alertent le risque est réel que les recettes actuelles soit diminuer jusqu'à 70% avec les règles européennes en vigueur. Ce serait un encouragement singulier au mode routier et un frein puissant aux politiques publiques de report modal. Il faut donc bien reprendre aujourd'hui, dès aujourd'hui, la question majeure du rééquilibrage de compétitivité des modes de transport durable par rapport au mode routier. Demain si la collectivité européenne d'Alsace réussi à mettre effectivement en place sa taxe sur le transport routier de marchandises. Elle montrera qu'il est possible d'agir sans que ce soit une catastrophe économique pour les transporteurs. Tous les exemples européens en attestent. Il faudra que la région Grand-Est puisse agir elle aussi sur le sillon lorrain de façon à éviter les dégâts de report et ces avancées en perspective indique assurément une voie qui sera nécessaire pour tout le réseau routier principal du pays. C'est ainsi, je crois que nous arriverons à plus de cohérence européenne en la matière. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à madame Nadège avait pour le groupe RDPI pour cinq minutes. rapporteure Madame la Ministre, mes chers collègues. Il y a une semaine nous débattions des réponses européennes à apporter aux récentes mesures protectionnistes américaines pour soutenir le développement de notre industrie verte. Afin de maintenir notre cap le zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050, j'ai pu rappeler à cette occasion au nom de mon groupe, la nécessité d'apporter une réponse forte on européen. Simplification de la procédure de des projets importants d'intérêt européen, assouplissement des règles sur les aides d'État. Réflexion sur la commande publique réorientation des financements vers les technologies propres formations aux métiers de demain. Voilà le chemin que nous empruntons ensemble ce nouveau projet de loi Dadu par la 36 position et la mise en conformité de plusieurs directives et règlements avec notre droit participent à cette construction collective. Les sénateurs du groupe RDPI voteront bien entendu ce texte. Car il permet de belles avancées en matière de droit du travail en matière d'égalité des droits et suite aux propos que j'ai tenu à l'instant, en soutien à notre ambition écologique. À l'issue des travaux menés par les députés et par nous en première lecture et je vous remercie nos rapporteurs 8 articles étaient conformes. 31 demeurait en discussion des compromis ont été trouvés. La commission mixte paritaire a été conclu conclusive et c'est toujours une satisfaction. La précision apportée au Sénat de la mention territoriale dans la transposition de la directive accessibilité à l'article 12 a été retenu, il s'agit de s'assurer d'une répartition territoriale équilibrée dans l'accès aux produits et services concernés sur l'article 9 qui transpose la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Celle-ci a été réécrite suite à sa suppression ici. Concernant l'article 5 bis qui prévoit un agrément préalable à l'exercice de la profession de prestataires de services sur actifs numériques une issue a été trouvée et plus Gobelins allemand je veux revenir sur 5 points majeurs du texte, le texte conduira je l'évoquais un instant à rendre plus accessible aux personnes en situation de handicap. Certains produits et services. Je pense au site internet à l'amélioration de l'accessibilité des distributeurs automatiques de billets et de titres de transport. Ou de bornes d'enregistrement automatique dans le domaine des transports publics ferroviaires. L'article 27 visent à renforcer les droits des voyageurs en situation de handicap et aux mobilité réduite À compter de juin 2023, les services régionaux devront leur apporter assistance à l'embarquement et au débarquement des trains et c'est du concret. En matière parental notre marge de j'aurais été allongée avec bonheur la durée du congé paternité. Mais aujourd'hui, lorsque le salarié s'absente dans ce cadre, cette absence n'est normalement pas comptabilisées dans le calcul de l'ancienneté. Alors que le congé maternité. De son côté est pris en compte dans son intégralité. Le projet de loi vient combler cette disparité en assimilant la durée d'absence à une période de travail effectif en matière de travail justement une obligation d'information sur les éléments essentiels de la relation de travail et créer dans le code du travail. Dans le domaine de la santé afin de protéger les consommateurs et les patients, les exigences à les exigences à respecter dans pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales vont être définies. Enfin dans le champ environnementale. L'article 26 vise à encourager un transport de marchandises plus écologique en conditionnant les taxes de circulation au nombre de kilomètres parcourus et à la quantité de dioxyde de carbone émise par les poids lourds cette modulation se substitue à celle prévue par la précédente version de la directive Eurovignette. Notre groupe fondamentalement attachés à la construction européenne et à ses exigences soutient ses nombreuses avancées. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant madame Corinne Ferré pour le groupe socialiste pour cinq minutes. Monsieur le Président Madame la Ministre monsieur le président de la commission, madame le rapporteur. Mes chers collègues. Notre droit s'enrichit régulièrement de dispositions décidées avec les autres États membres de l'Union européenne. Avec ce projet de loi, il s'agissait de transposer et de mettre en oeuvre plusieurs directives et règlements adoptés ces 3 dernières années, mais aussi de nous mettre en conformité. Sur la forme je souhaiterais rappeler que les délais accordés au Sénat pour l'examen de ce projet de loi ont été particulièrement contre une telle manière de procéder n'est pas acceptable dans une démocratie respectueuse des droits du Parlement, a fortiori pour un texte technique exigeant un temps d'expertise nécessaires à l'application des directives à transposer l'obligation voire l'urgence à légiférer pour adapter le droit interne au droit de l'Union européenne ne saurait justifier des délais particulièrement courts que nous a laissé le gouvernement. Pour le reste, ce texte est un peu fourre-tout avec sa trentaine d'articles portant sur des questions économiques et financières de santé publique ou encore de transport qui n'entrait pas moins de sujets importants et qui vont, pour certains dans le bon sens, comme en matière d'accessibilité des trains régionaux aux personnes en situation de handicap ou de meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et Il est à présent le fruit d'un compromis trouvé en commission mixte paritaire ce dont nous nous satisfaisons. Après cette CMP. Nous saluons l'amélioration porté à l'article 12 qui vient étendre les obligations issues de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation, la citoyenneté des personnes handicapées. Cet article habilite le gouvernement à transposer la directive du 17 avril 2019 relatives aux exigences en matière d'accessibilité applicable aux produits et services. Celle-ci vise notamment l'accessibilité des terminaux en libre-service terminaux de paiement guichet de banque automatique distributeurs automatiques de titre de transport. En pratique, on constate que l'accès à ces terminaux varie fortement selon les territoires considérés conformément au souhait du Sénat la répartition territoriale équilibrée des terminaux en libre-service sera garanti par la loi, de sorte que soit notamment préserver l'accès des services bancaires pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est une bonne chose, même si l'enjeu réside plus aujourd'hui dans le calendrier de mise en oeuvre de ces obligations par les opérateurs économiques que dans l'adoption la promulgation de ces nouvelles règles en droit interne au regard des retards constatés dans l'application de la loi de 2005, le gouvernement devra faire preuve de volontarisme dans un pays où 12 millions de personnes, relève d'une situation de handicap, l'absence d'une société pleinement inclusive constitue une anomalie, une atteinte de principes au principe d'égalité des droits et des chances. Nous sommes par ailleurs réservé sur l'article 8 qui habilite le gouvernement à transposer la directive dite c'est des de 2022 relatives à la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises. Rappelons que cet article avait été supprimé par le Sénat, puis rétabli par l'Assemblée nationale dans une version différente de la version d'origine certes désormais l'habilitation et plus encadré. Mais il est toujours contrariant de voir se multiplier les demandes d'habilitation à légiférer par ordonnances, d'autant plus en l'espèce lorsqu'il s'agit d'une opération allant au départ bien au-delà de la simple transposition en droit interne la directive c'est SRD avec cet enjeu particulier de la transparence des entreprises et du reporting de la durabilité nécessité selon-nous un travail approfondi. Ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'une étape importante du Pacte Vert européen dans le cadre duquel des choix déterminants vont devoir être effectués. Nous aurions donc préféré un vrai texte. Autrement dit, un projet de loin une procédure législative ordinaire permettant de débattre sereinement et de lever les questions restant en suspens. Malgré ces quelques réserves qui appellent notre vigilance. Le groupe socialiste, écologiste et républicain votera ce texte. Quand nous sommes avant tout des européennes et des européens convaincus. Je vous remercie. Merci cher collègue. Conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie de la santé, du travail des transports et de l'agriculture dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire modifié par l'amendement que nous avons adopté tout à l'heure du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Le projet de loi est adopté. Merci madame la ministre je vais suspendre quelques instants, le temps que. Monsieur Béchu et l'amabilité d'arriver.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement la procédure accélérée visant à ouvrir le tiers-financement à l'état ces établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. Ce texte est examiné selon la procédure de législation en commission prévu aux chapitres 14 bis du règlement du Sénat. La parole est à monsieur Christophe Béchu Ministre de la Transition écologique et la cohésion des territoires, vous avez la parole. Monsieur le ministre. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs Madame. La rapporteure. Eustache-Brinio. Transition écologique et cohésion des territoires. C'est très exactement ce dont il s'agit avec. Cette proposition de loi. Comment. Soutenir les élus locaux, en particulier en faisant en sorte de leur donner les moyens d'accélérer sur la rénovation des bâtiments publics dans un contexte et une équation que nous connaissons une urgence climatique de l'autre et des montants financiers qui sont colossaux. D'un autre côté. Notre pays comme. Toute l'Europe est engagé dans. Une stratégie de décarbonation dont nous connaissons les termes faire en sorte en 2030 d'avoir diminué nos émissions de gaz à effet de serre de 55% pour atteindre cet objectif, il faut jouer sur tous les leviers. L'énergie. Ça a été le cas. Avec. À la fois le projet de loi sur les énergies renouvelables qui a été voté, ça le sera quand celui sur le nucléaire, l'aura été de manière définitive. Jouer sur les infrastructures. Et là c'est la remise imminente du rapport du comité d'orientation des infrastructures et les efforts que nous allons avoir à faire, en particulier otite du ferroviaire pour la décarbonation. Et puis il y a un 3ème grand levier qui concerne la rénovation des bâtiments dans la rénovation des bâtiments, il y a 2 types de bâtiments. Les logements individuels le résidentiel, c'est environ deux tiers des émissions pour ça, il y a un dispositif perfectible améliorable MaPrimeRénov et qui a déjà permis d'engager un million et demi de rénovation et dont on va faire en sorte de continuer à améliorer la performance. Puis on a la partie publique, de la rénovation. Les bâtiments qui ne sont pas des bâtiments résidentiels, c'est un tiers des émissions. Et à l'intérieur de ça. On a une part considérable qui concerne les bâtiments publics, plus d'un tiers du parc tertiaire. Nous parlons de 400 millions de mètres carrés. Dans ces plus de 400 millions de mètres carrés, on en a environ 100 qui appartiennent à l'État. Et plus de 300 qui appartiennent aux collectivités locales et dans les 300 millions de mètres carrés qui appartiennent aux collectivités locales un mètre carré sur deux et scolaire. Écoles, collèges ou lycées. Et donc c'est pas seulement du Patrimoine dormant mais c'est du Patrimoine vivant dans lequel la transmission des savoirs et la préparation de la relève des futures générations se se fait. Cette proposition doit, elle vise à faire oeuvre. D'efficacité et d'exemplarité d'efficacité parce que si on ne rénove pas le parc public, on n'attendra pas nos objectifs et d'exemplarité parce que que l'état ou les élus locaux encouragent leurs concitoyens nos concitoyens à faire des efforts sur leurs propres Timone si on ne le fait pas sur le nôtre, ça pose une petite difficulté sur le caractère prescriptif de ce que nous disons. Le problème, il est assez simple, c'est quand on dit qu'il y a 400 millions de mètres carrés et qu'une partie significative de ce parc est à rénover et qu'on applique des ratios moyens des coups d'isolation des bâtiments. On arrive à des factures qui se chiffrent en centaines de milliards. Comment, dans le contexte des finances publiques que nous connaissons faire face. Les subventions et les crédits ont une limite. Même en ayant rajouté un fonds Vert doté de 2 milliards d'euros en ayant des crédits issus du plan de relance en ayant la déciles qui peut servir à une partie tout ça des tout ça des certificats d'économie d'énergie. Un fonds chaleur que vous avez majorée de 150 millions d'euros par rapport à la trajectoire et qui atteint 100, 120 millions d'euros. On est à 4 milliards si je prends la somme à financer et le montant des subventions j'ai évidemment Delta. L'idée. C'est donc de sortir du cadre. Et. De desserrer le frein à la rénovation des bâtiments publics qui est l'impossibilité de lisser les paiements et donc de se rembourser sur les économies d'énergie stratégique que beaucoup d'acteurs privés sont en train de déployer. La réalisation de travaux de rénovation énergétique serait. Dans le cadre du code de la commande publique. Possible avec un paiement différé, dans le cadre de marchés globaux de performance énergétique avec une dérogation spécifique. Qui ne serait pas la réhabilitation des partenariats public-privé mais qui serait bien un mode qui nous permettrait à la fois de conserver une exigence de gestion publique et un levier pour que les élus qu'ils veulent, ceux qui ne veulent pas. Se saisiront, pas de la faculté qui leur sera offerte avec le vote du texte puisse utiliser ce dispositif. En quelques mots. C'est bien l'idée. D'une autorisation pour une durée de 5 ans de conclure des contrats de performance énergétique. 5 ans, ça n'est pas la durée de réalisation des travaux d'amortissement. C'est la période pendant laquelle on peut contracter ce type de produit. Ça n'est pas un PPP parce qu'on peut faire un partenariat public-public. Par exemple en s'appuyant sur son intercommunalité sur la banque des territoires sur une sème une SPL ou un syndicat d'énergie et donc en ayant pas la difficulté de se demander quel est le niveau de profit ou de rentabilité du dispositif. Et ça n'est pas non plus un PPP parce que on ne délègue que le chantier par la gestion du bâtiment. Et donc on reste à l'exception de la délégation du chantier dans une maîtrise. Cette proposition de loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, elle a été adoptée à l'unanimité en commission des lois au Sénat et cette unanimité tiens. Au travail de votre rapporteur, que je tiens à saluer la sénatrice. Eustache-Brinio, notamment parce que les amendements qui ont été fait par le Sénat me semble apporter à la fois quelques garde-fous. Et quelques incitant supplémentaires dans le cadre du dispositif en particulier. En étendant le bénéfice de l'expérimentation aux actions de mutualisation des travaux de performance énergétique menée par les EPCI où les syndicats d'énergie, on est très clairement. Dans le fait d'aller lever une partie des freins que j'évoquais il y a quelques instants, mais. Dans le même temps. La simplification de la procédure de la vérification demander aux collectivités est cruciale parce qu'on sait que si le texte est trop lourd, les collectivités les plus petites ne s'en saisiront pas. Or ce sont sans doute elle. Qui ont les épargnes les plus contrainte et qui les rendent les plus. Loin de la possibilité sans ce type de dispositif de pouvoir avancer. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Je souhaite évidemment que ce texte fasse. L'objet du vote le plus large possible. Je veux simplement vous livrer en terminant ma conclusion avec 3 réflexions à haute voix. La première, c'est qu'en votant ce texte ne contraignant personne, on ajoute dans la boîte à outils de tous les élus de ce pays une possibilité d'avoir un mode de financement innovants sur quelques années qui nous permet de sortir de l'injonction de ne rien faire c'est ne pas réagir à l'action climatique et faire quelque chose c'est prendre le risque de se retrouver avec des montants de finances publiques qui sont complexes. Ah. Comblée, là on a une solution. Rationnelle qui s'inscrit dans la durée et qui apporte non seulement un bienfait immédiat pour le climat pour le pouvoir d'achat ou en tout cas pour les dépenses budgétaires des collectivités à moyen terme. Mais avec un bienfait particulier, ce sont les usagers de ces bâtiments parce qu'on raisonne comme si on était seulement en train de décarboner ou dépenser de l'argent dans une école il y a des enfants. Il y a des enseignants et la qualité de cours elle dépend aussi du niveau et de la chaleur qu'il peut y avoir dans le bâtiment de quand on leur a voté. Et c'est ce que je fais en temps masqué. Il faudra que les véhicules qui permettent de s'en saisir, de manière simple existe d'ingénierie. Of de prêts structurés dispositif permettant d'accompagner y compris les régions ou les départements qui déciderait de les accélérer sur leur territoire. Ce travail avec la banque des territoires. Il sera dans un mois. Capable de déboucher sur un programme qui sera si vous votez ce texte et s'il fait l'objet d'une CMP conclusive possible a proposé à tous les élus locaux de ce pays. Enfin et c'est là-dessus que je termine plus largement dans une année où nous allons avec l'AMF avec l'ADF avec l'ARF discuter de ce que sont les Budgets vers la manière de regarder comment par rapport aux dépenses qui sont à faire, il peut y avoir des soutiens de l'État qui peuvent être accrue sur ce qui est vertueux pour le climat ou pour la biodiversité. On est aussi dans cet exercice qui consiste à montrer ce qu'une dette verte qui consiste à investir de l'argent d'aujourd'hui pour éviter des dépenses plus élevées demain parce que le climat est un usurier et que l'inaction un coup qu'on n'est pas encore totalement capable de mesurer. Nous ferons. Oeuvre utile dans cette dimension également un immense merci pour votre attention. Monsieur le Ministre, la parole est maintenant Madame, Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteur de la commission des lois pour 7 minutes.

Il me revient désormais de vous présenter brièvement la proposition. La position de la commission des lois sur ce texte qui présente à première vue une forte dimension technique mais dont les enjeux sont considérables, aussi bien pour pour améliorer le confort des usagers et des agents du service public que pour réussir effectivement la transition énergétique de notre pays sans dérapages financiers. Pour rappel, et comme vous l'avez détaillé monsieur Ministre derrière l'utilité assez aride de cette proposition de loi se cache un dispositif somme toute assez simple, il s'agit de déroger à titre expérimental au code de la commande publique afin de permettre à l'État aux collectivités territoriales et à leur établissement public respectifs d'initier plus facilement des travaux de rénovation énergétique en différant le paiement de ces travaux de façon à ce que ces derniers puissent être financés par les économies d'énergie qui devrait entraîner le paiement initial des travaux est ainsi réalisé par un tiers, d'où le terme tiers-financement cette expérimentation représenterait ainsi un nouvel outil à la disposition de l'État et des collectivités territoriales. Confronté à l'engagement d'investissements colossaux au regard des objectifs particulièrement ambition ambitieux pardon de réduction de la commode consommation d'énergie des bâtiments publics que nous avons inscrit dans la loi une première fois dans la loi Grenelle 1 de 2009 puisse à nouveau dans la loi de 2008, la loi Elan. La loi Elan impose donc notamment une réduction de 60% de la consommation des finale des bâtiments publics d'ici 2050 par rapport à leur niveau de 2010. L'atteinte de ces objectifs bien évidemment louable représente néanmoins un défi collectif colossal tant les sommes sont importantes à mobiliser et qui pourraient apparaître démesuré. Vous l'avez rappelé monsieur ministre d'après les estimations qui nous ont été transmises il faudrait engager à minima. Près de 400 milliards d'euros pour procéder à la rénovation énergétique des 400 millions de mètres carrés détenue par les propriétaires publics pour la seule faire la seule sphère étatique les montants évoqués atteignent 80 milliards d'euros. Je n'ai donc évidemment pas été surprise de constater lors des auditions que nous avons menées. Et. Des mots que nous avons entendu l'incapacité d'atteindre ses objectifs sans mobilisation des ressources sans mobiliser des ressources supplémentaires dédiés à la mise à niveau du parc immobilier du secteur public selon les termes de la direction de de l'immobilier de l'État qui a pourtant déjà mobilisé beaucoup et tout près de 4 milliards d'euros à la rénovation énergétique de cécité administrative depuis 2019. Dans ce contexte. Évidemment par la hausse récente des coûts d'énergie. Le texte qui nous est proposé peut indéniablement représenter une solution pour aider l'ensemble des propriétaires publics à relever le défi de la transition énergétique, il ne fait aucun doute que cette expérimentation permettra à certains projets de voir le jour en bénéficiant d'un plan de financement adéquat. En aucun cas cependant ce texte peut être présenté comme évidemment mais tout le monde le sait, une solution miracle qui nous dédouaneraient de toute réflexion supplémentaire sur les moyens que que nous nous donnons pour achever la transition énergétique du secteur public. Nous avons vu cette expérimentation davantage comme un outil complémentaire pour favoriser cette transition qu'un remède indolore pour allonger alléger le budget des collectivités territoriales peinant à respecter leurs engagements en matière de rénovation énergétique. Il convient de rappeler que c'est pour de bonnes raisons que la jurisprudence constitutionnelle tout comme le droit commun de la commande publique encadre très strictement le recours au tiers-financement et au paiement différents différé auquel cette proposition de loi permettrait de déroger. En effet le tiers financeurs répercutera évidemment et nécessairement sur l'acheteur public. Le coût de l'avance de trésorerie que représente le paiement différé ce dispositif sera donc plus coûteux pour la public un financement classique qu'soit sur fonds propres ou par le biais d'emprunt bancaire s'être Marc m'apparaît d'autant plus fondée que l'ensemble des personnes que nous avons interrogées partagent le même constat selon lequel les économies d'énergie ne pourront pas compenser le coût total des travaux de rénovation. C'est une réalité. En outre, nous avons constaté que les conditions de passation de ces contrats inspiré des marchés de partenariats peuvent parfois parfois semblé assez lourde, ce qui risque de limiter fortement l'intérêt du dispositif pour certains propriétaires publics c'est pour se quoi. La commission des lois à apporter des modifications au texte transmis au Sénat afin de rendre plus accessible cette expérimentation tout en maintenant l'exigence de soutenabilité financière des projets notamment lorsque ceux-ci engagent plusieurs acheteurs publics dans ce cas la part supportée par chaque acteur public sera devra être clairement identifiés, préalablement à la signature du contrat. Dans l'objectif de favoriser les synergies locales, nous avons en outre étendu le dispositif expérimental aux établissements publics de coopération intercommunale et au syndicats d'énergie qui pourront prendre en charge comme l'autorise le code général des collectivités territoriales, les travaux de performance énergétique pour le compte de leurs membres en parallèle et en réponse aux réserves que nous avons évoqués, nous avons renforcé le suivi et l'évaluation de cette expérimentation afin d'une part que les dérogations au code de la commande publique soit pleinement justifiée. À l'issue d'un retour d'expérience du. Et d'autre part que les collectivités en difficulté puissent rapidement être identifiés et donc accompagné compte tenu de ces améliorations. Donc ils t'ont, qui ont été apportées à ce texte lors de l'examen en commission des lois. La commission s'est effectivement prononcé à l'unanimité en faveur de l'adoption de ce texte. Merci cher collègue. La parole est maintenant Madame Jocelyne Guidez pour le groupe Union centriste pour cinq minutes.

Monsieur le président. Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. La rénovation énergétique des bâtiments est indéniablement, l'une des principales solutions de maîtrise de la consommation d'énergie telle qu'signer aux personnes publiques dès 2009 et le de participation à la réduction de l'empreinte carbone. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans cette stratégie de rénovation énergétique des bâtiments publics, des différents acteurs, lesquels mettent en avant à juste titre une double nécessité d'exemplarité et d'atteinte de nos objectifs en la matière. En effet le Patrimoine immobilier du secteur public représente 400 millions de mètres carrés dont un peu plus de train des trois quarts sont détenus par les collectivités et le rétablissement, une évaluation des sommes nécessaires aux travaux de rénovation énergétique d'un tel parc. Excusez-moi. C'est comme ça. Se chiffrerait en plusieurs en centaines de milliards d'euros. C'est pour cela que la direction de l'immobilier de l'État évoque la nécessité d'une mobilisation de ressources supplémentaires. C'est là tout l'enjeu soulevé pour. C'est par cette PPL, le financement de ces travaux. En effet, ceux-ci peuvent représenter des sommes faramineuses pour les personnes publiques et particulièrement pour ce qui est des bâtiments scolaires, lesquels représentent la moitié de la surface totale des bâtiments publics, des collectivités locales. Ces propositions de loi nous amène à parler du tiers-financement comme solution à ce problème. Un mécanisme de facilitation permettant d'inclure un tiers dans le portage financier d'une rénovation. Le dispositif central de ce texte réside ainsi dans une expérimentation pour 5 ans d'une dérogation aux dispositions du code de la commande publique, lequel interdit actuellement tout paiement différé dans les marchés passés par l'État. Ces établissements publics, les collectivités leur établissement public et le regroupement. Cette dérogation vise les contrats de performance énergétique conclu sous la forme d'un marché global de performance pour la rénovation énergétique, ces contrats restent peu employé par les acheteurs publics on en dénombre seulement 380 sur les 15 dernières années. Il est donc nécessaire que les personnes publiques s'approprie mieux cet outil nous soutenons cette idée car c'est une solution pertinente. D'autant qu'elle consiste en une expérimentation. Ce qui nous permettra de procéder à une évaluation rigoureuse, éventuellement d'en corriger les défauts. Nous nous réjouissons des félicitations d'accès à cette expérimentation adopté en commission notamment l'extension du bénéfice de cette expérimentation à la prise en charge des travaux de rénovation énergétique par les EPCI et syndicats d'énergie pour le compte de leurs membres. J'en profite d'ailleurs pour saluer la qualité du travail mené en commission sous l'impulsion de notre rapporteur Jacqueline Eustache Brunoy les délais étaient contraints. Mais elle a su malgré tout apporté des améliorations l'assouplissement des conditions de mise en oeuvre a rapporté à l'article 1er bis est également. Bienvenu l'expérimentation pourra ainsi à devenir dès lors que le bilan préalable est au moins aussi favorables que les autres modes de passation, cet article a également le mérite d'accroître le degré de précision de l'étude de soutenabilité budgétaire ce qui contribuera à prévenir les situations de surendettement toutefois certaines interrogations subsistent comme le soulevé en commission notre collègue Françoise Gatel sur certaines entreprises proposant davantage du copier-coller que de l'justement au cas par cas, ainsi que sur la nature de la dette engendrée par les collectivités. La question reste en effet posée de savoir s'il faudra considérer cette dette comme une dette verte et le dispositif qu'il sera possible d'associer ou de mettre en place afin d'accompagner au mieux les causes les collectivités mais pas seulement dans leur effort de rénovation énergétique des bâtiments. Ce que nous appelons, je le crois, de tous nos. à ce stade, vous l'aurez compris, chers collègues, nous voterons en faveur de cette proposition de loi, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant madame la présidente Nathalie Delattre pour le groupe RDSE pour cinq minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la rapporteure Jacqueline mes chers collègues. Entre les records de chaleur régulièrement battu à des dates incongru puis les vagues de froid les déficits pluviométriques et l'augmentation du coût de l'énergie. Ces derniers mois, continue de souligner l'urgence climatique et l'impérieuse nécessité à agir pour tous, dont les pouvoirs publics. Les francs sont multiples, modes de production d'énergie, traitement des déchets, protection des espaces naturels adaptation de la mobilité et des transports. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui. Question de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est évidemment un enjeu de taille, puisque l'immobilier les constructions représentent dans notre pays, plus d'un tiers de la consommation d'énergie et près d'un quart des émissions de dioxyde de carbone. Et il va sans dire que les bâtiments publics qui tiennent une place considérable qu'il s'agisse des écoles, collèges, lycées, des hôpitaux et de l'ensemble des administrations. Nous partageons tristement chaque année le constat que les travaux de rénovation sont trop peu mises en oeuvre dans le secteur public. Pourtant il y a unanimité à vouloir s'engager dans de réelles politique publique de rénovation énergétique des bâtiments. Cette proposition de loi me paraît s'inscrire dans une dynamique attendue d'ailleurs pour toutes les lois, celle de de davantage de souplesse pour plus d'efficacité. De la souplesse car elle offre un nouvel outil, le recours au tiers-financement sans en supprimer d'autres. Il a été observé une trop faible utilisation des contrats de performance énergétique. Face, souvent à la difficulté que représentait l'investissement pour les collectivités territoriales et tout particulièrement pour les petites communes. Les règles de la commande publique sont contraignantes. Le plus souvent pour de bonnes raisons d'autant que l'usage des deniers publics doit être. Strictement encadrée. Ces motifs justifient donc d'interdire tout paiement différé dans les marchés passés par l'État, les établissements publics ou les collectivités territoriales. Toutefois cette contrainte ne doit pas conduire à ce que l'administration s'isole sans jeu de mots du reste de la société et ne l'accompagne. Pas dans ces défis fondamentaux l'introduction du tiers-financement pourrait donc permettre aux administrations, la réalisation de travaux d'envergure. Mais dans le coût serait lisser dans le temps. Je pense qu'il s'agit d'une option intéressante et dans son ensemble, le groupe RDSE souscrit à cette souplesse. joue. Souscrivons pardon d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un moyen imposer aux collectivités mais d'une nouvelle solution, laquelle s'ajoute aux autres déjà existantes. Cela étant, cher collègue. Il faudra demeurer vigilant. Comme nous devons l'être à chaque fois que nous assouplissant les règles d'utilisation de l'argent public. Heureusement, ce nouveau dispositif sera expérimental et pour une durée limitée à 5 ans. À l'issue de ce délai à notre charge d'observer si les collectivités se sont effectivement saisi de l'outil que nous créons et de veiller à ce qu'ils n'aient pas été perçu comme trop complexe pour être mise en oeuvre. Il faudra aussi nous assurer qu'en renonçant aux règles de la commande publique. Nous n'avons pas contribuer à générer de mauvaises pratiques ou de mauvaises dettes mauvaise parce que le remboursement ne serait pas si simple qu'annoncé. Mais aussi parce que les travaux de rénovation ne serait pas aussi efficace qu'espéré. Bref, le travail d'évaluation propre à chaque expérimentation devrait être fait le plus sérieusement possible sans quoi la pérennisation du dispositif ne pourra être acceptable le Sénat et la Chambre idéal pour ce faire, il reste que notre groupe est dans son ensemble favorable à la proposition de loi, nous le sommes d'autant plus au regard des améliorations apportées lors de l'examen en commission, madame la rapporteure. Nous vous soutenons madame la rapporteure pour rendre plus accessible. L'expérimentation en permettant notamment la prise en charge des travaux de performance énergétique par les EPCI et les syndicats d'énergie tout comme nous vous soutenons sur le renforcement de certains mécanismes de contrôle comme l'étude de soutenabilité budgétaire avec ces ajustements. opté devrait donc opte adopter un texte équilibré et le groupe RDSE s'en réjouit. Je vous remercie. Merci madame la présidente. La parole est maintenant Madame Valérie Boyer pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.

Nous achevons de travaux de cette semaine par l'examen d'une proposition de loi touchant de sujets pour lesquels notre assemblée et tout s'est toujours montrée très attentive, à savoir les finances des collectivités territoriales, bien évidemment et l'environnement. Ce texte de prime abord assez technique vise à ouvrir la procédure de tiers-financement aux entités publiques afin de permettre l'accélération des travaux de rénovation énergétique de près de 400 millions de mètres carrés de du bâti publique c'est quand même énorme. Cette accélération est effectivement indispensable, si nous souhaitons atteinte des objectifs de réduction de la consommation d'énergie d'énergie fixée depuis la loi sur le Grenelle de l'environnement de 2009. Cela d'autant plus que dans ce contexte économique et géopolitique actuelle. La maîtrise de ses consommations est devenue un enjeu crucial. Je n'ai certainement pas besoin de vous rappeler les difficultés que rencontrent certaines communes qui, confronté à la hausse abrupte du prix de l'énergie sont forcés de faire des choix très difficiles, d'ailleurs, des fois on y arrive même pas cette détresse, nous l'avons tous entendu dans nos échanges avec les élus locaux de nos territoires élus qui font un travail remarquable dans nos communes. Malgré un contexte de plus en plus difficile, notamment avec cette précarité énergétique qui les touchent comme elle a touché les français dans ce climat financier dégradé, il devenait d'autant plus difficile d'effectuer des investissements nécessaires au financement de rénovation et d'isolation pour ces mêmes communes souvent propriétaire d'un foncier abondant et vieillissant. Il faut dire que les outils juridiques actuels avait déjà montré leurs limites. Les contrats de performance énergétique. Relativement peu utilisé que ce soit sous la forme d'un marché global de performances ou d'un marché de partenariat de performance. Au final, seuls 383 contrat de ce type pur conclu entre 2007 et 2021. Un chiffre bien décevant au regard de l'ampleur du travail qui reste à faire. En réaction à cela. Le texte nous arrivons de l'Assemblée nationale. Poser d'assouplir l'ex-expérimentalement certaines règles de la commande publique afin de permettre la participation de tiers et donc de son privés comme cela a été très bien expliqué à ce travail de rénovation dans le cadre des marchés. Globaux de performance en contrepartie de versements ses talents dans la durée. Plus simple à concrétiser qu'un marché de partenariat et préservant la maîtrise d'ouvrage de personnes publiques ce dispositif contribuera à lever l'un des freins à l'investissement dans la rénovation énergétique. L'idée sous-jacente et naturellement de permettre. Aux économies générées par la rénovation énergétique d'équilibrer le coût inhérent au recours aux financements extérieurs. Cependant, comme l'a très justement relevé en commission notre rapporteur notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio et j'en profite pour la remercier de son travail important le dispositif proposé par ce texte évidemment n'est qu'un outil complémentaire auquel notre approche de la gestion ne saurait se limiter. Il n'a pas vocation à être systématique Zé et ne doit pas devenir une source de fragilisation des finances publiques locales d'autant plus qu'il est à ce stade plutôt difficile de quantifier l'ampleur réelle des économies qu'il saura susceptible de générer. In fine, et les choix de financement décisif se feront souvent directement en situation à l'échelon local, pour garantir une approche équilibrée de près de 10 amendement furent adoptés en commission. Ceux-ci permettent d'étendre le bénéfice de cette expérimentation aux EPCI au syndicats d'énergie mais affine également les exigences de soutenabilité budgétaire entourant celle-ci en effet, il est impératif que les contrats ainsi conclu constitue bien un outil de financement au moins aussi favorables que ceux dont dispose déjà les collectivités. Il en va. D'une bonne logique je dirais mais surtout du bon usage des deniers publics, sur lequel nous devons être absolument intraitable quand nous travaillons sur un chantier d'une telle ampleur. Enfin, même si à titre personnel j'ai. C'est-à-dire que la remise d'un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue par ce texte ne constituera pas un frein. Elle sera sans doute l'occasion de dresser un bilan qui informera non seulement la question de l'éventuel maintien de ce dispositif, mais aussi les tendances gouvernant l'évolution de l'effort de rénovation du bâti public en France et à titre personnel aussi, je me réjouis qu'on ait un rapport d'évaluation parce que ça nous est souvent refusé pourtant c'est extrêmement important d'avoir à la fois des études d'impact qui ne manque cruellement je faire référence au texte sur les retraites par exemple ou des rapports qui nous sont refusés, c'est essentiel qu'on puisse en avoir. D'ici là. Pour en revenir à ce texte là et pour permettre d'améliorer le pilotage du dispositif pendant la durée d'expérimentation. La commission a également proposé qu'il fasse l'objet d'un suivi régulier par le gouvernement et fasse l'objet d'un rapport de mi-parcours, donc on voit bien tout l'intérêt du contrôle qui est le nôtre. compte tenu de toutes les améliorations que le Sénat a apporté et du travail qui a été fait en commission au Sénat. Notre groupe est disposée à voter le texte tel qu'il ressort bien entendu des travaux de la commission, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant au président Claude Malhuret, pour le groupe. Les indépendants pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la décarbonation du bâti public est un défi majeur pour notre pays. Nous savons que notre parc immobilier se déprécie peu à peu, jusqu'à bientôt pour certains. Pour certaines de ces partis ne plus répondre aux normes en vigueur. Vous avez parlé, Monsieur le ministre de la rénovation de 4 à 500 millions de mètres détenue par l'État et les collectivités. Les investissements nécessaires sont colossaux. Les enjeux immenses et les travaux pharaoniques. Il devient chaque jour plus urgent d'accompagner les élus pour que teindre les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de rénovation énergétique des objectifs d'une ampleur considérable qui nous engage à apporter des outils à la hauteur. Ce texte permet à l'État et à ses établissements publics, mais aussi aux collectivités et à leurs groupements de recourir au tiers-financement. Il s'agit donc de lisser dans le temps les investissements réalisés dans le cadre de contrats de performance énergétique. Le dispositif a été encadré et sécurisé par les apports du Sénat. Il est désormais adapté aux réalités des territoires ruraux en permettant aux EPCI d'assurer les travaux pour le compte des communes. Cette expérimentation puisqu'il s'agit bien d'un essai temporaire est une carte supplémentaire dans le jeu des élus locaux. Une nouvelle carte qui permettra non seulement de compléter les outils existants d'alléger le budget des collectivités territoriales, mais aussi d'expérimenter une solution plus souples. Nous en tirerons par la suite tous les enseignements nécessaires grâce au bilan des élus pionniers. Mes chers collègues, la philosophie générale du texte que nous examinons aujourd'hui va dans le bon sens. Le soutien apporté au dispositif par les associations d'élus était un bon indicateur. Nous poursuivons dans le même sens. L'adoption de cette proposition de loi à l'Assemblée puis au Sénat apporte de nouvelles solutions concrètes aux élus. Elle les accompagne dans l'atteinte de nos objectifs environnementaux par une expérimentation innovante. Nous pouvons nous en féliciter. Parmi les différents dispositifs destinés aux élus locaux. Le Fonds Vert va dans le bon sens l'autorisation à recourir au tiers-financement aussi nous en tirerons toutes les conclusions avant d'envisager son éventuelle généralisation. Si nous voulons réduire l'empreinte carbone nationale, nous devons mobiliser toutes les solutions dont nous disposons. Le contexte actuel nous rappelle l'urgence des réponses à apporter. Il est particulièrement important d'envoyer un signal de souplesse en ce moment pour faciliter le déclenchement des projets locaux. Les investissements ont parfois été ralentie et les ambitions revues à la baisse en cette période d'inflation énergétique. Les factures que reçoivent les élus ces derniers mois, souligne le caractère vétuste de certains bâtiments. Nous ne pouvons plus accepter de conserver des passoires thermiques dans le parc immobilier public. Par l'adoption de ce texte, le Parlement donne le coup d'envoi de nombreux projets de grande ampleur. C'est une bonne nouvelle pour l'environnement, ça l'est tout autant pour nos territoires et pour le dynamisme de nos communes. Le groupe des Indépendants Monsieur le Ministre accueille donc favorablement cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci monsieur le président. La parole est maintenant monsieur Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste pour cinq minutes.

C'est le président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. La Cour des comptes a autant le dernier noter la cohérence et le risque d'inefficacité des mesures gouvernementales destinées à améliorer leur prête environnemental des bâtiments. Ce même rapport après que le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire constitue en France, la première chose de consommation d'énergie. 44%. La politique de rénovation énergétique des bâtiments à laquelle l'État a consacré plusieurs réformes législatives au cours de la dernière décennie est un outil majeur bien sûr pour la mise en oeuvre de la stratégie bas-carbone et de l'accentuation de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce constat d'octobre dernier. N'est pas nouveau la rénovation énergétique oui est un outil majeur au service de la transition écologique. Notre groupe alerte depuis bien longtemps sur ces problématiques de passoires thermiques et les charges que cela fait peser sur de nombreux foyers modestes. Pour autant, les bâtiments publics sont loin d'être épargnée par la surconsommation d'énergie des bâtiments publics de l'État et des collectivités locales sont responsables dans les communes de 76% de la consommation énergétique à Marseille. La municipalité a établi qu'une école publique sur 3 de la ville était en situation préoccupante. Certaines écoles dépasse largement les seuils de consommation énergétique moyenne avec une surconsommation. Estimée à 20.000 mégawatts par an, soit la consommation électrique annuelle totale d'une ville de 7000 habitants. L'effort sur les écoles par exemple a trop longtemps été repoussé les diverses échéance se rapprochant les factures continuent de s'envoler le coût du filet de sécurité si utile et des rénovations éventuel ne doit pas être pris à la légère retrouve dans le cas du Patrimoine public. La double peine que vivent les foyers. Le coût de la dette climatique est bien trop nocif pour notre société. Vous l'avez rappelé. Monsieur le Ministre, c'est un usurier et l'urgence est là. La présente, proposition de loi que nous avons étudié en commission tente de répondre à la problématique du coût très élevé des travaux souvent nécessaire et propose une expérimentation pour 5 ans d'aménagement du droit de la commande publique particulièrement sur le paiement différé. Conscient de l'attente des collectivités et favorable à l'accélération de la transition énergétique et des bâtiments publics. Notre groupe est en faveur de cette expérimentation, mais certaines interrogations demeurent. En effet le risque d'une captation par le secteur privé d'une grande partie de la rentabilité des activités économiques engendrées par les économies d'énergie à la faveur ou sous la forme de privatisation de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux et de leur financement et réel des femmes PPP partenariat public-privé. Souvent hélas était accompagné d'abus de la part des partenaires. Privés. Le marché de la rénovation thermique représentant une source de profit importante pour les entreprises ils semble judicieux de bien s'interroger sur tout dispositif financier simplifiant le recours au privé plutôt qu'à des acteurs publics par la mise en oeuvre de mécanismes encadrant la dépense publique l'inertie des dernières décennies a déjà un coup, il convient de s'assurer qu'il ne soit pas encore amplifié. Au delà de cette expérimentation, c'est bien la question du financement de la transition énergétique qui se pose. Et je salue le constat de notre rapporteur sur le sujet cette PPL n'apporte qu'un dispositif complémentaire bienvenue mais qui ne peut représenter l'unique solution pour réussir la transition énergétique du secteur public. Surtout que le tiers-financement ne doit pas être favorisée de façon systématique en raison des surcoûts qui l'entraîne. J'espère que beaucoup sur ces bancs sont d'accord sur le principe de pollueur payeur et défendraient une taxation des entreprises les plus polluantes qui pourrait mieux alimenter le budget de MaPrimeRénov'ou de toute autre dispositif pour aider la rénovation énergétique des logements des particuliers. L'expérimentation proposées dans ce texte reste une bonne idée la réelle ambition d'évaluation de cette expérimentation voulue par notre commission est indispensable au vu des sommes qui pourraient être engagées. L'objectif de réduction de 60% de la consommation énergétique des bâtiments publics d'ici 2050 ne peut se faire sur des mécanismes d'accompagnement des mécanismes si possible pérenne et les moins coûteux. Cette expérimentation va permettent de dresser le bilan des mécanismes qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Notre chambre des territoires connaît bien les difficultés auxquelles sont confrontés les collectivités. La crise énergétique et les discussions sur le filet de sécurité ont montré que ces difficultés étaient présentes partout en milieu rural comme en milieu urbain dans les petites collectivités comme dans celle de grande taille. Cette loi n'apportera qu'une partie très limitée de réponse aux ambitions qui doivent être les nôtres de rénovation thermique et ne permettra pas à elle seule de les atteindre. Mais elle va dans le bon sens. Notre groupe la votera mais il restera attentif aux possibles dérives des marchés de rénovation et il continuera à travailler sur ce sujet prioritaire, notamment au travers de la commission d'enquête sur la rénovation énergétique des logements que notre groupe a initié avec notre président Guillaume Gontard, en tant que rapporteur. Merci, merci, cher collègue, la parole est maintenant madame Nadège avait pour le groupe RDPI pour cinq minutes. Merci monsieur le président, madame la rapporteure. Monsieur le Ministre, chers collègues, la loi de 2018 portant évolution du logement, de l'Aménagement et du numérique a imposé une réduction de 60% de la. Consommation d'énergie finale des bâtiments publics d'ici à 2050 par rapport à leur niveau de 2010 alors que le secteur du bâtiment génère 23% des émissions de gaz à effet de serre, l'attente de la neutralité carbone en 2005 en compte pour les bâtiments publics de plus de 1000 m2 représente un défi majeur à relever. Ce cap que nous nous fixons est ambitieux et surtout nécessaire nos objectifs ronde impératif un effort massif et continu notamment budgétaire afin de soutenir la rénovation énergétique du parc immobilier. La presse a pu à ce propos, parler de chantier du siècle et c'est très juste. Vous l'avez rappelé. Monsieur le Ministre, nous parlons de 400 millions de mètres carrés de bâtiments publics et pour un coût total de plusieurs milliards d'euros de rénovation. C'est d'ailleurs. Partant de ce constat que notre groupe a souhaité user de son droit de tirage en 2023 pour la création d'une mission d'information sur le bâti scolaire à l'épreuve de la transition écologique et nous nous intéressons spécifiquement avec mes 22 collègue aux écoles au collège et au lycée qui couvre la moitié du parc tertiaire des collectivités territoriales. 12 millions d'élèves, ils sont accueillis chaque année. Face à ces enjeux qui touchent à notre quotidien de nombreux leviers doivent être activé afin de pouvoir bénéficier d'expertise juridique et technique de qualité et pour faciliter et diversifier les sources et les modalités de financement. Le dispositif innovant dont nous discutons aujourd'hui se veut justement une réponse pertinente qui s'inscrit pleinement dans ce cadre d'action déposée en novembre 2022 par la présidente, Aurore Bergé, le groupe Renaissance. La proposition de loi ton conformément aux objectifs de massification précité à encourager. Faciliter le recours des personnes publiques au contrat de performance énergétique encore trop peu utilisé pour ce faire et pour lever les freins à l'investissement qui résulte du coût élevé que représentent les travaux le texte que nous nous apprêtons à deux d'adopter pardon vient déroger sous forme expérimentale pour une durée de 5 ans au code de la commande publique. Il vise ainsi à permettre à l'État aux collectivités territoriales et à leur établissement public respectifs d'engager plus facilement des travaux de rénovation énergétique en différents leurs paiements. Il s'agit ni plus ni moins de lisser le coût de la rénovation en faisant part porté par un tiers le paiement immédiat des travaux, d'où le terme de termes de tiers-financement cela permettra un remboursement progressif sous forme de loyer annuel en partie réalisé grâce aux économies d'énergie générée. Il s'agit bien bel et bien d'un nouvel outil au service de la transition énergétique. va être qu'il devra être évoluer un dispositif complémentaire parmi d'autres. Il vient ainsi s'ajouter, d'une part au partenariat public-privé qui permet aussi le tiers financièrement mais qui, en matière de rénovation énergétique ne sont quasiment jamais utilisé par les collectivités territoriales et d'autre part aux marchés globaux de performance pour les élus locaux le tiers-financement leur permettra de conserver la maîtrise d'ouvrage et de contractualiser sur une forme qui intégrera le financement et la réalisation des travaux de bout-en-bout. Madame la rapporteure. La commission a adopté dans le cadre de la. Procédure de législation en commission 10 amendements. L'objectif, Fax, faciliter l'accès à l'expérimentation de ce régime hybride, tout en maintenant une forte exigence en matière de soutenabilité financière des projets développés en la matière. Monsieur le Ministre vous avez par ailleurs demandé à la banque des territoires d'élaborer un outil qui permettrait aux communes de bénéficier d'une aide en matière d'ingénierie et de s'assurer de la confiance dans le tiers-financement le groupe RDPI se prononcera en faveur de ce texte et souhaite que ce dispositif soit opérationnel dès cet été, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant monsieur Jean-Yves Le Leconte pour le groupe socialiste pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre. Madame la présidente madame la rapporteure, mes chers collègues. Grenelle de l'environnement. Accord de Paris. Loi élan à chaque fois des engagements et. Finalement, la nécessité de se concentrer sur la rénovation énergétique selon le principe que la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas. Depuis. Là. Les objectifs de l'Union européenne en matière de. De réduction. Des des des émissions carbone en particulier la volonté d'être neutre en 2050 et l'objectif de moins 55% en 2030, conduit aujourd'hui les le le le l'Union européenne a engagé un un trilogue sur. En particulier la mise en oeuvre d'un marché carbone pour le bâtiment et transports qui est susceptible, s'il n'y a pas de rénovation de coûter encore plus cher aux utilisateurs et à ceux qui utilisent de l'énergie pour les bâtiments. C'est la raison pour laquelle. Il est absolument important de répondre à cette exigence. Surtout après ce que nous avons vécu depuis un an. Ce coup de tonnerre sur ce qui a remis en cause les habitudes européennes en matière d'énergie, c'est-à-dire l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine qui finalement met en évidence la dépendance de nos économies aux combustibles fossiles et a renchéri significativement la facture de énergétique de l'ensemble des Français mais aussi des collectivités. C'est la raison pour laquelle. Il est absolument indispensable de trouver des des des des solutions en particulier pour un, un parc immobilier public, ça a été dit, de 400 millions de mètres carrés et dont l'estimation dans votre rapport, madame la rapporteure. C'est à peu près 400. Milliards, 400 milliards, plus de 20 points de PIB autour de 20 points de PIB de coups. Si nous devions mettre cela en place d'un seul coup, c'est la raison pour laquelle c'est absolument indispensable de trouver des outils. Même si on peut aussi s'interroger sur finalement l'adéquation des moyens même des nouveaux moyens aux enjeux qui nous attendent. En tout état de cause. Même si ça ne résoudra pas tout, compte tenu des enjeux et des et, des et des besoins de financement. Le principe de, de la proposition de loi qui est d'introduire une expérimentation visant à inclure un tiers dans le portage financier et technique d'une rénovation énergétique de bâtiments de rejoint ainsi aux articles du code de la commande publique qui encadre les investissements et dépenses publiques est intéressant le tiers et d'investissement et. Du commanditaire. L'État, une collectivité territoriale ou un établissement public, le remboursement de l'avance et des intérêts, compte tenu des besoins urgents signalés. Nous ne pouvons que saluer ce texte qui est une avancée intéressante. Il faudra se simplement veiller à à quelques éléments d'abord à ceux qui ne favorise pas les, les gros maître d'oeuvre. Ceux qui disposent d'ingénierie financière au détriment. Des petits artisans et des PME qui participe grandement à la vitalité de nos territoires. Ça c'est une première inquiétude, la capacité de financement finalement des acteurs dans dans ce domaine et il faudrait être particulièrement vigilante. Deuxièmement, comme beaucoup d'autres intervenants dans cette DG. Bien entendu avec des collectivités qui sont. Monsieur le Ministre moins aidé par l'État avec des collectivités qui subissent elles aussi une précarité financière compte tenu de la situation et des coûts de l'énergie. Actuellement les risques. D'accumulation de d'engagements financiers ne serait-ce qu'avec ces nouveaux outils mérite d'être largement surveillée. Nous avons vu l'effet des PPP sur un certain nombre de collectivités, mais aussi sur, par exemple le ministère de la justice et il ne faudrait pas revenir sur des outils qui conduisent aux mêmes dérives il est particulièrement bienvenue d'avoir un, un suivi et de faire ceci de manière expérimentale. Nous avons besoin de ces outils mais nous ne pouvons pas faire comme avec les les PPP et ses réserves étant tout en regrettant bien entendu que l'Union européenne et l'État ne mettent pas plus de moyens pour. Aller dans cette direction, au niveau européen des de la rénovation énergétique des bâtiments publics. C'est en soutenant mais avec une certaine vigilance que le groupe socialiste, écologique et républicain se prononcera en faveur de cette proposition de loi. Merci, cher collègue, la parole est enfin madame Michelle Gréaume pour le groupe CRCE pour cinq minutes. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, chers collègues, je tiens à saluer la volonté du gouvernement via son groupe à l'Assemblée de mettre au coeur des débats la transition écologique. Ce sujet est important et nous devons y porter une attention particulière tant les enjeux sont forts et dans chacune de nos actions et de nos décisions ont un impact sur l'environnement sur nos vies et celles des générations futures. Aujourd'hui, nous devons nous prononcer sur le financement des travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics de l'État. Des établissements publics et de nos collectivités territoriales par Chair financeurs. Celle-ci est un sujet complexe et très coûteux. Chers collègues, vous le savez on le voit au quotidien la précarité énergétique et réel sujet et beaucoup de ménages subissent au quotidien leur logement. Mal isolé. L'objectif, 1er de répondre aux enjeux de transition écologique. Pour cela, nos bâtiments publics doivent être exemplaires. Ils s'étendent sur près de 400 millions de mètres carrés aux trois quarts appartiennent aux collectivités territoriales. Chaque année l'énergie pour chauffer des bâtiments des équipements ou des bâtiments représentent de 6%. De la consommation finale d'énergie du pays. Ah, bâtiments publics sur 2 est un établissement scolaire si l'école et mal isolés. La spirale négative se met en place, non seulement le coût de fonctionnement pèsent sur le budget, mais aux causes. D'autres contrats tels que maladie professeur absent canicule des fermetures d'écoles, ces 400 millions de mètres carrés qu'il faut rénover. Nous reconnaissons que cette proposition de loi apparaît comme un outil pour accompagner la rénovation énergétique, notamment pour permettre à certaines communes surtout en ruralité de pouvoir lever les freins sur des investissements. Nous serons très attentifs au suivi et à l'évaluation de la mise en oeuvre de cette loi. Cependant, nous restons très dubitatif sur l'effet levier espéré par cette dernière. La rénovation énergétique. Quand on veut se conformer aux normes actuelles et bénéficier des meilleurs au standard nécessite d'autres dépenses qui ne peuvent être dissociées de ces travaux. Mise aux normes des réseaux électriques sécurité anti-incendie normes PMR, sans compter les imprévus. C'est toute la structure du bâtiment qui doit être prise en compte pour réaliser de réelles économies d'énergie. Il faut également prendre en compte les coûts financiers qu'appliquent les rénovations. En effet, cela nécessite de grands moyens humains dans un contexte où le secteur du bâtiment subi une importante pénurie de main-d'oeuvre. Des formations sont nécessaires pour répondre aux défis actuels de rénovation certains ouvriers ne dipose pas de ces diplômes et d'autres n'ont pas les moyens d'envoyer les équipes en formation. Concernant les TPE-PME seront les sacrifiés de cette proposition de loi au profit des grandes boîtes du BTP qui ont les moyens d'avancer les fonds pour des travaux. La crise sanitaire a mis en grande difficulté, les petites entreprises. De plus, quatre élus sur 10 affirment qu'ils n'accéléreront pas leurs projets de transition écologique au motif qu'ils n'ont pas les moyens de les mettre en oeuvre les collectivités sous contrat de faire des choix dans un moment de crise sociale énergétique qui met en difficulté les finances locales. Contrairement à l'État. Ces dernières doivent présenter un budget équilibré. Les économies d'énergie espéré par cette proposition de loi. Ah si, que l'impact sur leur vie. Ne semble pas être réellement mesurée. Les les collectivités sans visibilité. Et sa sécurité vis-à-vis de leurs dettes. Il ne faut pas non plus que 7 expirant expérimentation. Ah l'État à se désengager auprès des collectivités. Ah, véritable plan de rénovation pour les bâtiments publics surtout scolaire porté par l'État est indispensable. Pour toutes les raisons évoquées. Le groupe CRCE s'abstiendront sur cette proposition de loi lorsque les premières évaluations apparaîtront sur le sujet. Nous serons attentifs et nous ajusteront notre position si nécessaire. Merci. Si. Merci cher collègue. Je vais mettre aux voix, la proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l'état à ces établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. La proposition de loi est adopté. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, je vais lever la séance prochaine séance mercredi 1er mars à 15h pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est levée.